La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 18 juillet 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observations ? Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Charles Ceccaldi-Raynaud, qui fut sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2004,

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République. Mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 86 du règlement au scrutin secret pour l'élection à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences et la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote. Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Pour le cas du vote pour un titulaire assorti du nom de son suppléant, la radiation de l'un des deux noms entraîne la nullité du vote pour l'autre. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je remercie nos collègues Mmes Jacky Deromedi et Patricia Schillinger, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Les juges à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat. Je déclare ouvert le scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République. Il sera clos dans une demi-heure. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

Outre l'article relatif à l'aéroport, ceux qui portent sur l'indivision foncière constituent une réforme importante, sur laquelle les Polynésiens fondent beaucoup d'espoir. C'est cet espoir qui s'est exprimé mercredi dernier, lorsque j'ai inauguré le tribunal foncier de Papeete. Pour le Sénat, ces dispositions ne sont pas inconnues, puisque votre assemblée les a déjà adoptées, lors de l'examen du texte devenu la loi du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Comme vous le savez, ces éléments ont été écartés par le Conseil constitutionnel, par sa décision du 27 juin dernier, pour des motifs uniquement procéduraux.

Ce soutien gouvernemental est d'autant plus naturel que les dispositions relatives à l'indivision ont été construites grâce à un travail très minutieux accompli par la Chancellerie avec le Gouvernement de la Polynésie et sa direction des affaires foncières, les magistrats présents sur place, les avocats, les notaires, les géomètres, les généalogistes même, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs locaux intéressés. Je ne reviendrai pas sur le détail de ces dispositions ; votre votre rapporteur, M. Darnaud, vous les rappellera certainement. Je souhaiterais m'arrêter ici un instant sur la méthode que nous avons employée. Cette méthode montre que la justice sait s'adapter aux réalités et aux besoins des justiciables, partout en France, dans l'Hexagone comme dans les outre-mer. Nous avons, pour cela, inversé la logique qui a longtemps prévalu concernant les outre-mer. Souvent, trop souvent, la République a préféré plaquer un modèle unique sur l'ensemble des territoires et des populations, alors que la diversité des situations exigeait, au contraire, que l'on trouve des solutions un peu différenciées, approchant au plus près les réalités que nous avions à traiter. Des progrès ont été accomplis ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire pour inverser cette logique et acquérir ce « réflexe outre-mer » que promeut ma collègue Annick Girardin. La manière d'aborder la question foncière dans les outre-mer, et singulièrement en Polynésie, illustre cette volonté qui est la nôtre de changer de logiciel. Sur l'indivision, je ne vous apprendrai rien ce phénomène a été particulièrement bien analysé dans le rapport de 2016 de la délégation sénatoriale aux outre-mer, coordonné par votre collègue Thani Mohamed Soilihi. Ce rapport constitue le travail de référence sur cette question. Il y était fait le constat d'un état généralisé d'indivision transgénérationnelle, rendant difficile toute utilisation ou disposition de la terre. Pour la Polynésie française, le rapport avait mis en avant les particularités historiques, culturelles, juridiques propres à ce territoire, qui conduisent à des situations totalement inextricables, avec, souvent, un nombre très important de co-indivisaires- plus encore que dans les autres outre-mer -, pouvant atteindre plusieurs centaines de personnes dans certains cas. Parmi ces spécificités, celle relevant de la géographie n'est pas la moindre

particularités, l'absence fréquente d'adresses précises empêchant de localiser correctement les ayants droit, de les attraire à la cause, de les assigner et de leur signifier les décisions, le nombre important de contentieux de revendication de terres sur le fondement de la prescription acquisitive, le recours quasiment systématique aux partages judiciaires, ce qui allonge considérablement les délais de procédure, et, enfin, l'absence de représentation obligatoire par avocat en première instance.

Cette réalité est bien identifiée par le Gouvernement, ainsi qu'en témoigne la mise en oeuvre récente de moyens inédits. En cela, je poursuis et intensifie une action dont les premiers éléments ont été mis en place par mes prédécesseurs, Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas. Une importante avancée résulte de la mise en place, le 1 décembre 2017, d'un tribunal foncier à Papeete, fonctionnant sur le mode de l'échevinage et doté de moyens humains et matériels propres. propres. Il est désormais installé dans un bâtiment neuf adapté à ses missions et à l'accueil des justiciables. Sa création et son fonctionnement constituent une réussite, comme j'ai pu le constater sur place, auprès aussi bien des magistrats que des justiciables. Le stock des dossiers, ainsi que leur durée moyenne de traitement, ont été notablement réduits, ce qui favorise l'apaisement des situations. Les Polynésiens, désormais dotés d'un tribunal dédié aux affaires de terre, se sont pleinement approprié ce dispositif, ainsi qu'en l'augmentation récente du nombre des requêtes déposées. Par ailleurs, afin de soutenir l'action de la direction des affaires foncières de Polynésie, la pratique du salariat d'avocats dédiés au contentieux foncier par cette direction a pu être consacrée dans la loi organique de juillet dernier. les moyens ainsi mis en place devaient impérativement être accompagnés de mesures relatives au fond du droit des indivisions et des successions. C'était une revendication ancienne des autorités polynésiennes et des magistrats exerçant sur place, revendication qui n'avait jamais pu aboutir compte tenu de la complexité des situations. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Cette question avait déjà été mise en avant par les parlementaires de Polynésie, en particulier la sénatrice Lana Tetuanui, que je salue ici chaleureusement, lors de la discussion, en 2018, de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, à laquelle le Gouvernement a apporté son soutien. Ce texte est désormais entré en vigueur à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lors des débats sur cette proposition de loi, en 2018, la situation propre à la Polynésie française a été mise en évidence. Il fallait aller plus loin pour apporter des réponses adaptées,

Il était indispensable d'approfondir davantage la réflexion afin de trouver un équilibre entre la nécessité de mettre en place des outils pragmatiques et efficaces pour lutter contre l'indivision et le respect des droits fondamentaux, tels que le droit de propriété, les droits de la défense de l'ensemble des héritiers indivisaires et les droits des conjoints survivants. C'est ainsi que, le 4 janvier 2018, lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale en outre-mer, je m'étais engagée devant vous, à ce que la question de l'indivision en Polynésie française soit expertisée sérieusement et rapidement par la Chancellerie afin d'aboutir à des solutions concrètes. Cet engagement a été tenu avec la création d'un groupe de travail, lancé en 2018 et piloté par mon cabinet, le Gouvernement de la Polynésie et les parlementaires élus dans ce territoire, dont je salue l'investissement personnel. Ce groupe de travail a réuni pendant plusieurs mois des représentants de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction générale de l'outre-mer et de la direction des affaires foncières de Polynésie, mais également des magistrats, des avocats et des notaires de Papeete. Cette étroite collaboration a été fructueuse, puisqu'elle a débouché, en quelques mois, sur la rédaction de plusieurs dispositions, que vous avez votées par voie d'amendements lors de l'examen du projet de loi sur la Polynésie française et qui sont reprises dans dans cette proposition de loi. Ce texte comporte ainsi des dispositifs innovants, dont certains sont l'adaptation de ceux adoptés dans le cadre de la loi du 27 décembre 2018 pour les autres outre-mer. Je pense par exemple à l'attribution préférentielle, à l'omission d'héritier et au partage amiable à une majorité qualifiée. D'autres dispositions visent à répondre à la situation spécifique de la Polynésie française, avec notamment le partage par souche et le droit de retour légal des frères et soeurs. La rédaction concernant le partage par souche témoigne vraiment du souci commun du Gouvernement de la République et du Gouvernement de la Polynésie française d'avancer ensemble, puisque, si l'ossature du dispositif que nous proposons d'inscrire dans la loi est de la compétence de l'État, il est renvoyé, pour le détail de son organisation, à la loi du pays, s'agissant notamment de règles de procédure civile qui relèvent de la compétence propre de la Polynésie française. Lors d'une réunion de travail tenue sur place, dimanche dernier, il y a donc quarante-huit heures, avec le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, et plusieurs de ses ministres, nous avons évoqué ces questions et passé en revue toutes les actions engagées par son gouvernement pour s'attaquer à l'indivision. Je dois avouer que j'ai été très impressionnée par l'ampleur de l'action qui est menée sur place, avec le souci constant de tenir compte des réalités de chaque île, la situation pouvant varier d'un archipel à l'autre. C'est donc un texte important qui vous est soumis aujourd'hui. J'ajouterai que cette proposition de loi comporte également une disposition relative au contrat de concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'État en Polynésie française. Vous avez d'ailleurs déjà examiné et voté ce dispositif,

et votre engagement pour nos compatriotes polynésiens, soutenu par le Gouvernement, nous permettent d'espérer un vote conforme de votre assemblée et une entrée en vigueur très rapide de ces textes, moins d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel. C'est vraiment important pour la Polynésie. Je peux vous assurer que, dans tous les archipels, des îles Marquises aux Australes, en passant par les îles de la Société et les Tuamotu-Gambier, on attend ce texte.

en déposant sa proposition de loi, le 1er juillet dernier, notre collègue député Guillaume Vuilletet a souhaité réagir à la décision de non-conformité partielle rendue par le Conseil constitutionnel le 27 juin 2019 concernant la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi ordinaire par le Premier ministre en même temps que de la loi organique adoptée le même jour, a en effet estimé que certains articles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions initiales ; il a prononcé une censure d'office sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a voulu rétablir rapidement les articles censurés en déposant cette proposition de loi. C'est une initiative louable, qui a cependant été conduite de manière quelque peu précipitée et incomplète. Absolument ! Huit articles ont été censurés comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Or seuls six d'entre eux ont été repris dans la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Ont été laissées de côté les dispositions relatives aux crématoriums et à la dépénalisation du stationnement payant, pourtant attendues par les Polynésiens. Je vous rappelle que, faute de base légale, la crémation des corps ne peut être effectuée en Polynésie française. L'article censuré avait été introduit par le Gouvernement à la demande de l'Assemblée de la Polynésie française. Quant à la dépénalisation du stationnement payant opérée par la loi Maptam de 2014, elle empiète sur une compétence locale en matière de réglementation pénale et routière. Là encore, c'est le Gouvernement qui avait souhaité faire sortir la Polynésie du champ du dispositif. Ces deux sujets méritaient donc d'être repris dans la proposition de loi initiale, mais, passé le dépôt du texte, il est devenu inopportun et impossible de les rétablir : inopportun pour ne pas retarder une adoption conforme et permettre une entrée en vigueur rapide du texte, et, surtout, impossible en raison des règles de recevabilité de l'article 45 de la Constitution. Je précise que des amendements visant à rétablir ces articles ont été déposés à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Ils ont été déclarés « cavaliers législatifs » à chaque fois, dans la droite ligne de la décision du 27 juin 2019 du Conseil constitutionnel.

puissent être éventuellement reprises dans le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui sera présenté devant notre assemblée au mois d'octobre prochain. Le texte qui nous est soumis comprend cinq articles visant à faciliter la gestion et la sortie de l'indivision foncière et un article précisant le cadre des concessions des aérodromes d'État. Le Sénat a déjà eu l'occasion de les examiner et de les adopter. Les dispositions relatives aux indivisions successorales s'inspirent, pour l'essentiel, des recommandations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer. L'article 1 vise notamment à adapter aux spécificités polynésiennes, en particulier l'ancienneté des successions, la condition de résidence exigée du conjoint survivant ou d'un héritier copropriétaire pour bénéficier de l'attribution préférentielle d'une propriété en application de l'article 831-2 du code civil. L'article 2 prévoit, quant à lui, un dispositif dérogatoire du droit commun permettant le retour à la famille du défunt sans descendant de la totalité des biens immobiliers qu'il détenait en indivision avec celle-ci. L'article 3 a pour objet d'empêcher la remise en cause d'un partage judiciaire par un héritier omis. L'article 4 tend à prévoir un dispositif dérogatoire et temporaire favorisant les sorties d'indivision jusqu'au 31 décembre 2028, en permettant le partage des biens immobiliers indivis sur l'initiative du ou des des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis. L'article 5 institue une expérimentation, jusqu'au 31 décembre 2028, du partage par souche, tel qu'il est opéré par la cour d'appel de Papeete, en interprétant de manière extensive la notion de représentation de l'article 827 du code civil. Enfin, l'article 6 de la proposition de loi précise le cadre juridique dans lequel l'État peut concéder l'exploitation d'un aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française, en prévoyant la création d'une société dans laquelle la Polynésie pourrait être associée à sa demande. Tous ces articles avaient été introduits par le Sénat, en commission ou en séance, dans la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Ils reprennent à l'identique les rédactions issues du texte élaboré le 7 mai 2019 par la commission mixte paritaire et approuvé par les deux chambres. La seule modification, apportée par l'Assemblée nationale, a été la simplification du titre initial. En cohérence avec ses précédents travaux et afin de permettre, comme chacun le souhaite,

Il n'est pas question pour moi de m'étendre aujourd'hui sur le contenu de cette proposition de loi, puisque nous avons déjà examiné et voté ces dispositions spécifiques à la Polynésie française en matière de gestion du foncier en matière de gestion du foncier et de plateformes aéroportuaires relevant de la compétence de l'État en Polynésie française. Il s'agit bien de deux sujets d'envergure pour le développement économique et durable de ma collectivité, dont l'urgence était signalée par les autorités du pays.

En effet, certaines dispositions des deux lois se rapportant au statut d'autonomie de la Polynésie française adoptées en mai dernier ont été censurées.

Polynésiens, portant sur notre contribution à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation. C'était, hélas, prévisible à la lecture de l'avis du Conseil d'État du 29 novembre 2018. Cette disposition est donc déclassée en loi ordinaire : dont acte. Ainsi, force est de constater que la rédaction actuelle de l'article 74 de la Constitution ne nous permet pas de conférer de valeur organique à de telles dispositions, qui sont pourtant fondamentales pour nous, en Polynésie. En conséquence, il m'appartiendra, lors de la révision de nos institutions, de solliciter une modification de l'article 74 de la Constitution pour y intégrer au mieux la « reconnaissance « reconnaissance particulière de l'État à l'égard de la Polynésie française » afin de tenir compte de nos intérêts propres au sein de la République et de permettre la sanctuarisation de la dette dite « nucléaire Comptez sur moi, le moment venu, pour « revendiquer » l'inscription de cette assise forte et pérenne dans l'article 74 de notre Constitution, pour l'avenir de mon territoire.

Je découvre une jurisprudence renforcée et sévère du Conseil constitutionnel, dont découle un droit d'amendement fortement encadré et limité. Néanmoins, le Gouvernement central s'est aussitôt engagé à reprendre en partie ces dispositions et à les représenter le bon vecteur législatif. Ainsi, cette proposition de loi reprend six articles tels qu'ils avaient été adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il s'agit, en premier lieu, des cinq articles relatifs à la gestion et la sortie de l'indivision, qui adaptent tout particulièrement les règles en matière d'indivision successorale aux spécificités polynésiennes, avec un dispositif d'attribution préférentielle, un retour à la famille du défunt des biens immobiliers qu'il détenait en indivision, des droits spécifiques pour l'héritier omis et un partage possible par souche. Ces dispositions répondent parfaitement à la problématique polynésienne et s'inspirent fortement des recommandations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer.

En second lieu, le sixième article de cette proposition de loi reprend le cadre juridique dans lequel l'État peut concéder l'exploitation de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, qui avait été introduit au Sénat par amendement du Gouvernement et qui répond à une demande pressante et légitime des autorités du pays. Je comprends parfaitement l'urgence à légiférer dans ces deux domaines, mais je ne peux que regretter que, dans cette

Quoi qu'il en soit, je ne manquerai pas de représenter ces dispositions manquantes, avec d'autres mesures générales d'adaptation à la Polynésie française

Mes chers collègues, il est quinze heures cinq. Je déclare clos le scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République.

En effet, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre de cette loi ordinaire en même temps que de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, a estimé que certaines dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte initial. Il a ainsi prononcé une censure d'office sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a voulu rétablir rapidement les articles censurés en déposant cette proposition de loi.

Je déplore, tout comme notre rapporteur Mathieu Darnaud, que les dispositions relatives aux crématoriums et à la dépénalisation du stationnement payant aient été laissées de côté, alors que ces deux sujets méritaient d'y être traités. Faute de base légale, la crémation des corps ne peut être effectuée en Polynésie française, ce qui oblige les familles qui souhaitent y recourir à entreprendre des voyages onéreux en Nouvelle-Zélande. Quant à la dépénalisation du stationnement payant, opérée par la loi de 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, elle empiète sur une compétence locale en matière de réglementation pénale et routière. Néanmoins, je me félicite que la proposition de loi reprenne, dans les mêmes termes, les articles censurés par le Conseil constitutionnel qui permettaient d'adapter les règles en matière d'indivisions successorales aux spécificités polynésiennes, en particulier l'ancienneté des successions. Il s'agit des dispositifs d'attribution préférentielle, de retour à la famille du défunt des biens immobiliers qu'il détenait en indivision avec celle-ci, des droits de l'héritier omis, de la sortie d'indivision et du partage par souche. Ces dispositions s'inspirent, pour l'essentiel, des recommandations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer. La délégation avait mis en avant le caractère particulièrement complexe de la question foncière en Polynésie française, où « les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d'indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre à cinq générations et alimentent l'abondant contentieux des " affaires de terre Je me réjouis également que la proposition de loi reprenne un article précisant le cadre juridique dans lequel l'État peut concéder l'exploitation d'un aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française. Cette disposition prévoit que l'État peut imposer au concessionnaire- à la demande de la Polynésie française -de créer une société ad hoc associant l'opérateur économique qui dispose du pouvoir de direction et la Polynésie française. Madame la ministre, mes chers collègues, les élus polynésiens ne souhaitent pas que l'adoption de ce texte soit retardée. En effet, ces dispositions sont attendues de longue date. Par cohérence avec les travaux antérieurs et soucieux de permettre une entrée en vigueur rapide, le groupe Les Indépendants, même s'il considère qu'il aurait été opportun d'insérer dans le texte initial les deux dispositions relatives aux crématoriums et à la dépénalisation du stationnement payant, votera à l'unanimité cette proposition de loi.

portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et ordinaire portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, mon groupe avait déposé des amendements identiques à ceux de nos collègues polynésiens, Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey,

M. le rapporteur et moi-même étions les coauteurs, ces amendements avaient pour objet de faciliter la sortie de l'indivision, laquelle stérilise une grande partie du foncier disponible en Polynésie, celui-ci étant, rappelons-le, déjà rare. Nous avions, en accord avec les parlementaires polynésiens, fait le choix de les retirer de l'examen de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dont j'étais rapporteur, afin de les redéposer sur les textes précités. Cependant, le Conseil constitutionnel, saisi du projet de loi organique, a considéré que l'introduction de ces amendements dans le projet de loi ordinaire méconnaissait l'article 45 de notre Constitution, qui prévoit l'irrecevabilité d'amendements ne présentant aucun lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

cause. Elles prévoyaient l'attribution préférentielle du bien d'habitation à un héritier l'ayant occupé de façon continue, paisible et publique pendant dix années, sans exiger que l'habitation ait été effective au jour du décès. Elles permettaient également d'instaurer un droit de retour légal des frères et soeurs pour les biens en indivision reçus de leurs ascendants. Elles consacraient la possibilité de procéder à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est impossible. Elles adaptaient le dispositif issu de la loi du 27 décembre 2018 visant à établir un partage amiable des successions à une majorité de plus de la moitié des indivisaires. Enfin, elles permettaient d'exclure, pour l'héritier omis, l'annulation du partage, afin d'éviter une remise en cause trop importante des partages jugés, d'autant que ces derniers interviennent souvent au terme de procédures très longues et très coûteuses. Dans sa décision du 27 juin 2019, le Conseil constitutionnel a également censuré une disposition, introduite par le Gouvernement au Sénat, visant à encadrer la concession d'aéroports polynésiens. Le présent texte remédie à ce contretemps. Les dispositions qu'il contient sont très attendues par les Polynésiens. Celles qui sont relatives à la problématique foncière permettront le règlement des successions dans le respect des intérêts des indivisaires et de débloquer les politiques d'aménagement sur place. Les autres dispositions, notamment celles qui vont permettre d'encadrer la concession d'aéroports polynésiens, sont également attendues par nos compatriotes du Pacifique. Le groupe La République En Marche

la présente proposition de loi reprend des dispositions que nous avions déjà votées, en avril dernier, lors de l'examen des projets de loi sur la Polynésie française, adoptés par le Sénat à l'unanimité. La censure du Conseil constitutionnel, dont ont parlé les orateurs précédents, nous amène aujourd'hui à évoquer de nouveau la situation particulière de la Polynésie française, et plus largement des outre-mer, en matière d'indivision successorale, mais

Alors que vous avez, madame la garde des sceaux, inauguré la semaine dernière le tribunal foncier de Papeete, entité judiciaire unique en son genre, nous intervenons dans l'urgence afin de faciliter le traitement des contentieux juridiques en

Une autre cause historique ne doit surtout pas être oubliée : les méfaits de la période coloniale, qui a marqué la chair et l'esprit des Polynésiens, toujours habités par la peur de perdre leurs terres. La moitié des terres polynésiennes seraient aujourd'hui en situation d'indivision, avec un droit de propriété exercé à plusieurs en attente d'un partage, rendu complexe par le faible taux de démarches à l'amiable, qui amène un engorgement des tribunaux,

Créer un tribunal foncier ne suffit pas ; il faut donner les moyens aux juges polynésiens de résoudre les situations locales, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Notre groupe approuve l'adaptation du droit commun aux caractéristiques du pays en permettant d'alléger les conditions de partage et d'attribution préférentielle de biens, de donner aux frères et soeurs d'un défunt un droit de retour total des biens immobiliers en indivision, sauf usufruit légal du conjoint, de limiter les remises en question des décisions de justice et de recourir plus souvent au partage par souche. De telles mesures tendent aussi à reconnaître la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete, rejetée jusqu'à présent par la Cour de cassation. L'article relatif à la concession aéroportuaire devrait, quant à lui, inciter à relancer la procédure d'appel d'offres pour l'aéroport de Tahiti-Faa'a, attendue depuis longtemps. Tout en respectant l'indépendance du pouvoir politique polynésien, nous souhaitons, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, encourager le Gouvernement et le Parlement à légiférer plus régulièrement et plus naturellement sur les outre-mer pour permettre le bon fonctionnement de leurs institutions, mais aussi de la vie quotidienne des citoyens. Comme vous avez raison ! Nous appelons cependant à la prudence, car il ne doit pas seulement s'agir de consacrer à main levée des dispositions pour ces territoires. Encore faut-il en évaluer l'efficacité et l'impact sur les réalités locales,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, bien sûr,

qui conduit à réduire le volume de la production législative. L'histoire nous montre exactement le contraire ! Je regrette profondément cet état de choses.

que s'est-il passé ? À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, voilà que des députés, bien inspirés, ont décidé de faire une proposition de loi.

la Constitution de la République française : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement, en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de

Cela a été dit, il s'agit d'un texte spécifique, qui reprend sans modification des dispositions censurées le 27 juin dernier par le Conseil constitutionnel en tant que « cavaliers législatifs Je remarque que nous avions déjà discuté l'année dernière d'une proposition de loi portant sur l'indivision successorale en outre-mer. Sans doute serait-il d'ailleurs plus efficace et pertinent de travailler à un texte traitant globalement sur ces questions, plutôt que de légiférer au coup par coup, au gré des décisions du Conseil constitutionnel. La question est ainsi déjà largement balisée. Le rapport d'information de juin 2016 de la délégation sénatoriale aux outre-mer soulignait que l'indivision successorale et, plus largement, les incertitudes liées au droit foncier

Toutefois, il est aussi admis qu'en outre-mer la coutume joue un rôle important dans la régulation des rapports sociaux, ce dont l'État doit bien sûr tenir compte. Il ne serait ni aisé ni même peut-être souhaitable de vouloir aligner de façon stricte et abstraite les règles patrimoniales sur celles qui s'appliquent en métropole. En matière patrimoniale, française se caractérise par la fréquence de l'indivision transgénérationnelle- les successions ouvertes ne sont pas refermées, même après le décès des héritiers -, la succession se reportant sur la génération suivante, et ainsi de suite. Cette particularité peut avoir pour conséquence de rendre difficile toute utilisation de la terre et, bien souvent, les demandes de partage doivent être réglées par voie judiciaire, ce qui ne facilite évidemment pas les rapports sociaux et le bon usage du foncier et encombre les tribunaux. La proposition de loi apporte, dans une certaine mesure, des réponses à ces difficultés. Ainsi, l'article 1 permet à un héritier ayant occupé un bien pendant une durée de dix ans d'en bénéficier, même si l'occupation n'était pas effective au jour du décès. L'article 2 prévoit le retour, en l'absence de descendants, des biens à la famille du défunt. L'article 3 permet l'attribution d'une part à un héritier omis, sans remise en cause d'un partage déjà intervenu.

dans quelle mesure ce genre de questions est-il traité par les autorités locales, éventuellement par le biais d'une loi du pays ? Pour le dire d'une autre manière, si l'on comprend bien que les questions relatives à l'état des personnes relèvent de la compétence de l'État, quel peut être le rôle de la collectivité dans ce domaine ? La proposition de loi comporte également un dernier article relatif aux conditions d'exploitation d'un aérodrome situé en Polynésie relevant de la compétence de l'État. En pratique, celui-ci pourra, dans le cadre d'une concession, imposer la création d'une société associant les autorités polynésiennes.

Il constitue l'aboutissement d'un travail patient, dont les Polynésiens méritent aujourd'hui de voir les fruits. Ces dispositions portent principalement sur deux sujets : l'aéroport de Tahiti-Faa'a, d'abord, mais surtout la question de l'indivision successorale, qui pèse sur le quotidien de nos concitoyens en Polynésie. L'indivision successorale est un mécanisme bien connu de droit civil des biens qui permet de maintenir l'unité d'un bien ou d'un ensemble de biens après la mort de son propriétaire. Or les territoires ultramarins présentent des caractéristiques spécifiques, qui peuvent faire de l'indivision un véritable problème structurel. Celle-ci « bloque », dans une indétermination très inconfortable, une bonne partie du foncier local et conduit à une judiciarisation massive des successions. successions. Plus grave encore, les indivisions les plus anciennes peuvent donner naissance à des situations tout à fait inextricables, où beaucoup d'indivisaires sont inconnus ou injoignables.

Ce même texte avait également fait l'objet d'un amendement de notre collègue Lana Tetuanui, qui tendait à permettre le partage d'un bien par souche lorsque le partage par tête était impossible. d'ores et déjà, à prendre en compte un certain nombre des spécificités de la situation des indivisions polynésiennes. Le choix final avait été de retirer de ce texte les dispositions relatives à la Polynésie. Ce retrait s'était fait en accord avec le Gouvernement et les représentants du territoire ; il a permis de les inclure par la suite dans les deux projets de loi consacrés spécifiquement à ce territoire que nous avons examinés au printemps. Malheureusement, les sages du Conseil constitutionnel ont jugé que ces dispositions relatives à l'indivision, ainsi qu'un certain nombre d'autres dispositions, portant sur le cadre du fonctionnement de l'aéroport d'État de Tahiti-Faa'a, l'exploitation des crématoriums et la dépénalisation du stationnement payant, étaient des cavaliers législatifs. Elles ont donc logiquement censurées, pour des raisons de simple procédure, contre l'avis du Gouvernement. Cependant, la volonté obstinée de traiter durablement cette question a repris le dessus. Notre collègue député Guillaume Vuilletet s'est aussitôt mobilisé pour déposer la présente proposition de loi, qui constituera un véhicule législatif incontestable pour ces mesures. Venons-en à son contenu. Il porte la marque du Sénat, puisque ses articles 1 à 5 sont largement issus des travaux

facilitent le retour du bien à la famille du défunt, sécurisent les partages déjà intervenus et assouplissent les conditions de partage des biens indivis pour une dizaine d'années. En cela, ils se rapprochent des dispositions déjà en vigueur dans d'autres territoires ultramarins. En outre, l'article 5 du texte comprend un dispositif expérimental de partage par souche qui devrait permettre de tester sur place une pratique qui était déjà mise en oeuvre par les juges de première instance, mais souffrait d'un risque de cassation systématique. Il s'agit ici à la fois d'adapter le droit des successions aux conditions locales et de permettre un bon fonctionnement du service public de la justice. Nous ne pouvons évidemment que saluer cet usage de l'expérimentation. L'article 6, quant à lui, précise les conditions juridiques d'exploitation de l'aéroport principal du territoire et ne pose pas de problème particulier. Tout au plus pourrait-on regretter que les auteurs de la proposition de loi n'aient pas jugé bon d'y inclure également les dispositions censurées relatives aux crématoriums et au stationnement payant. compte tenu des circonstances, nous reconnaissons volontiers qu'une adoption conforme du texte issu de l'Assemblée nationale paraît aujourd'hui opportune, afin d'offrir dès que possible aux habitants de la Polynésie française les outils juridiques dont ils ont besoin pour résoudre ces questions délicates.

Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République : Nombre de votants : 258 Suffrages exprimés : 244 Majorité absolue des suffrages exprimés : 123

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, suppléante au poste de juge titulaire que vous m'aviez fait l'honneur de me confier, 244 voix. Ces candidates ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elles sont proclamées juges à la Cour de justice de la République.

de justice de la République. Je vais donner lecture de la formule du serment. Je prierai Mme la juge titulaire, puis Mmes les juges suppléantes, de bien vouloir se lever à l'appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d'être prêté devant lui.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a débouché, le 11 juillet dernier, sur un accord avec l'Assemblée nationale pour donner vie à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace. Cette nouvelle collectivité est le fruit d'une volonté forte des élus locaux, au premier rang desquels les présidents des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ainsi que celui de la région Grand Est, de redonner naissance à l'Alsace, dissoute lors du découpage des nouvelles grandes régions. Les négociations avec le Gouvernement ont abouti à l'adoption d'une déclaration commune, signée à Matignon le 29 octobre dernier, qui a servi de base à l'élaboration du projet de loi soumis au Parlement. Ainsi, la réunification des deux départements donne naissance à la Collectivité européenne d'Alsace, la CEA, qui est avant tout un département. Afin d'en faire plus qu'un simple département, mais moins qu'une collectivité à part entière et autonome, comme certains le revendiquaient, le projet de loi introduit certaines compétences nouvelles spécifiquement liées aux particularismes alsaciens, comme la coopération transfrontalière, le bilinguisme et la gestion du trafic routier. routier. Lors de la première lecture, le Sénat, après des débats houleux, avait souhaité aller beaucoup plus loin afin de donner à l'Alsace les véritables moyens de sa différenciation et d'offrir aux autres départements frontaliers la possibilité d'expérimenter. L'Assemblée nationale a préféré revenir à une version plus proche de l'accord signé à Matignon, tout en préservant des avancées significatives introduites par le Sénat. Ainsi, le texte issu de la CMP reprend les apports du Sénat concernant

effet, si l'accord ne retient pas toutes les garanties introduites par le Sénat, notamment l'introduction dans la base de calcul des dépenses d'entretien courantes inscrites au contrat de plan État-région, l'Assemblée nationale a accepté que l'éventuelle ne vienne pas en déduction des compensations financières. C'est tout de même une avancée significative. Je pense surtout à la neutralisation des conséquences, pour la Collectivité européenne d'Alsace, des engagements pris par l'État à l'égard de la société concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a maintenu diverses autres dispositions ajoutées par le Sénat, comme la possibilité pour l'État de déléguer la gestion des actions relevant du Fonds social européen, la création d'un conseil de développement, cher à notre collègue Guy-Dominique Kennel, et la possibilité de créer des chaînes de télévision locale, souhaitée par notre

Les travaux du Sénat, amplifiés par ceux de l'Assemblée nationale, ont permis d'aboutir à un accord tout à fait acceptable qui donne plus de contenu à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace qu'initialement prévu. Le Sénat a pleinement Le Sénat a pleinement rempli son rôle de chambre des territoires en écoutant le « désir d'Alsace » relayé par nos collègues sénateurs alsaciens, que je souhaite sincèrement remercier pour leurs éclairages, leurs conseils et leurs encouragements. Le pragmatisme du Sénat a surtout permis de sécuriser les effets du transfert de ces nouvelles compétences et d'alerter sur les difficultés à venir dans leur mise en oeuvre ce texte nous a donné un avant-goût des futurs débats sur le droit à la différenciation, montrant que l'attachement de chaque élu à son territoire justifie à ses yeux des particularités législatives. Enfin, comme le dit un bon proverbe alsacien, « la moitié d'un oeuf vaut mieux qu'une coquille entière ». Je vous invite à faire vôtre ce sage dicton et à adopter le compromis obtenu en commission mixte paritaire,

je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. En effet, ce texte est emblématique de la relation nouvelle que le Gouvernement souhaite promouvoir entre l'État et les collectivités territoriales, fondée sur les principes de confiance et de responsabilité. La contribution constructive des deux chambres à l'élaboration du projet de loi est par conséquent essentielle. Elle est le gage de la pleine participation du Parlement à la mise en oeuvre de la nouvelle méthode que nous avons l'ambition de fonder. Selon cette approche, l'action sur les territoires doit être le fruit d'une coproduction entre l'ensemble des acteurs. L'État assume, dans ce cadre, un double rôle de garant de la cohésion des territoires et de catalyseur du développement local. l'État assume la mission de faciliter l'expression des atouts de chaque territoire, en reconnaissant ses spécificités. C'est ce que nous avons pu démontrer, depuis l'engagement des travaux de concertation, en janvier 2018, pour répondre au « désir d'Alsace » que vient d'évoquer Mme la rapporteur.

Pour illustrer mon propos, je reviendrai très succinctement sur les conditions d'émergence de ce projet de loi. Il importe d'abord de rappeler que ce dernier est attendu par les acteurs locaux depuis l'échec du référendum de 2013 sur la collectivité territoriale unique d'Alsace et la création, en 2015, de la région Grand Est. C'est la raison pour laquelle le préfet de région s'est vu confier une mission de concertation. M. Jean-Luc Marx l'a remplie avec beaucoup d'intelligence et d'équilibre. Je voulais, à cette tribune, l'en remercier. Au terme de nombreux échanges avec les acteurs locaux et avec mes collègues du Gouvernement Élisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, une déclaration commune engageant le Gouvernement, les deux conseils départementaux ainsi que la région Grand Est a été signée le 29 octobre 2018. octobre 2018. Elle prévoit une réponse appropriée pour l'Alsace et trouve une partie de sa traduction dans le projet de loi que vous examinez. Ainsi, la création de la Collectivité européenne d'Alsace se matérialise par plusieurs étapes. étapes. Les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin seront regroupés en un seul au 1 janvier 2021, après que le décret du 27 février dernier a formellement procédé à ce regroupement. l'ajout, par la loi, de compétences particulières en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de transports. Enfin viendra le développement des politiques culturelles, économiques ou sportives dont les orientations étaient fixées dans la déclaration commune. font l'objet d'un travail approfondi avec les services déconcentrés de l'État et les autres niveaux de collectivités concernées ; elles se traduiront, pour la plupart, par des actes réglementaires. Je pense par exemple à la constitution d'un pôle d'excellence en matière de plurilinguisme et, plus prosaïquement, à la perspective de plaques minéralogiques alsaciennes. projet de loi est donc une composante centrale du dispositif que nous avons envisagé pour l'Alsace. Il s'attache à donner à l'Alsace des compétences suffisamment justifiées par des spécificités alsaciennes pour que le cadre constitutionnel actuel permette de les attribuer de façon pérenne et, bien sûr, circonscrite à ce territoire. Ainsi, au 1 janvier 2021, la Collectivité européenne d'Alsace exercera le socle classique des compétences départementales, auquel s'ajouteront quatre principales compétences. de compétences en matière transfrontalière : la collectivité aura la capacité d'organiser l'action collective, à travers un schéma de coopération transfrontalière. En parfaite cohérence avec la stratégie régionale, ce schéma pourra décliner un volet opérationnel sur les projets structurants. La CEA pourra ainsi se voir déléguer des compétences par l'État, la région ou des EPCI. deuxième lieu, des compétences en matière de bilinguisme afin de renforcer ce vecteur culturel et ce facteur de mobilité professionnelle que constitue la langue régionale, entendue ici, conformément aux conventions en usage, comme la langue allemande. Plusieurs leviers ont été identifiés : l'amélioration de l'attractivité des conditions d'embauche des enseignants d'allemand recrutés par le ministère de l'éducation nationale la possibilité, pour la Collectivité européenne d'Alsace, de recruter des intervenants afin de permettre l'enseignement de la langue au-delà des heures réglementaires, en complémentarité avec les programmes nationaux

territoire, la CEA animera et coordonnera l'action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. des compétences en matière d'infrastructures routières. Le projet de loi acte le transfert de la gestion et de l'exploitation des routes nationales et des autoroutes non concédées situées en Alsace. Si elle le souhaite, la Collectivité européenne d'Alsace pourra lever sur ces voies des ressources spécifiques

Les modalités de droit commun ont été rétablies pour le transfert des agents intervenant sur les routes, de manière à éviter de pénaliser la Collectivité européenne d'Alsace en cas de mouvements de personnel à la veille du transfert. Le principe de délégation des intercommunalités à la CEA a été maintenu. La création d'un conseil de développement a été retenue. Enfin, la référence faite au FSE est restée en l'état j'ai pu dire au banc qu'elle doit être considérée comme une invitation à poursuivre le travail engagé sur le guichet unique d'accompagnement des porteurs de projet. Vous l'aurez compris, le texte qui est soumis à votre approbation aujourd'hui est clairement le résultat d'un travail législatif constructif sur le fond, tout en demeurant dans l'esprit de la déclaration de Matignon, c'est-à-dire dans le cadre des orientations dessinées par le Gouvernement et les collectivités territoriales. Avant de conclure, je souhaite dire, une fois encore, que ce texte est une démonstration de bon augure de ce que le Gouvernement, le Parlement et les collectivités territoriales peuvent, chacun dans son rôle, répondre aux attentes de nos concitoyens et servir l'intérêt général. Je voudrais en ce sens remercier les acteurs territoriaux qui ont su oeuvrer pour que les conditions soient réunies pour la réussite de ce texte, au premier rang desquels figurent Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, et Jean Rottner, président de la région Grand Est. Je voudrais enfin saluer le travail de la commission des lois de son président, Philippe Bas, et de la rapporteur, Agnès Canayer, qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce processus législatif. Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui est soumis à votre approbation a été enrichi par le Parlement tout en restant équilibré. Il vient répondre favorablement à une volonté et à une ambition pour l'Alsace. C'est un jalon important de la politique menée pour les

Les divergences sur le texte entre les deux chambres étaient peu nombreuses, ce qui nous a permis d'atteindre un consensus rapidement. Il restera néanmoins un goût de déception globale, tant le champ des possibles induit par le sujet s'est finalement réduit. Je pense Je pense particulièrement aux potentielles avancées que le Sénat avait envisagées, mais qui ont finalement été rejetées par l'Assemblée nationale et le Gouvernement, ne laissant que peu de place à la réflexion positive. Ce texte a néanmoins le mérite d'exister et représente le fruit de l'aboutissement de plusieurs années d'échanges à tous les niveaux. Toutefois, il ne reflète que bien peu les attentes et les besoins des Alsaciens. Ce « désir d'Alsace », revendication positive, a été identifié par le préfet Marx dans son rapport. Loin d'évoquer l'aigreur d'un territoire replié sur lui-même, a entendu souligner ses particularités pour fonder, par une voie originale, un projet politique d'avenir, ancré dans les préoccupations économico-aménagistes de l'époque et profondément européen. Bien sûr, nous n'étions pas dupes de l'ambition politique de laisser renaître un ensemble institutionnel local qu'une politique récente avait, sans compromis possible, fait disparaître. Nous n'étions pas dupes non plus des difficultés d'explorer des voies du droit novatrices, dont les balisages habituels laissent peu de place à l'audace, malgré le consensus supposé de la démarche. de cette marge de manoeuvre réduite, nous avons néanmoins tenu à affirmer cette singularité territoriale, notamment en ce qui concerne le nom. Il était en effet important de conserver l'appellation de Collectivité européenne d'Alsace, qui, dès le début du processus, avait été retenue pour désigner le produit de cette initiative politique. Nous nous sommes inscrits, en tant que législateurs, dans les compétences qui nous sont reconnues en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution ainsi acté la variation d'une dénomination qui traduit ses particularités. En effet, aux côtés des collectivités territoriales de droit commun- communes, départements et régions -, dont le régime est caractérisé par une grande unité, le droit reconnaît des voies institutionnelles plus différenciées, destinées à permettre l'incarnation institutionnelle de réalités sociales particulières. La différenciation du nom au sein d'une catégorie de collectivité territoriale de droit commun constitue une expérience inédite. La différence du spectre de compétences de la Collectivité européenne d'Alsace au regard des départements classiques est manifeste. L'absence de reconnaissance de son caractère singulier par une appellation dédiée aurait constitué un manquement. J'en viens aux compétences. Certes, la solution d'une collectivité départementale a pour elle sa relative simplicité, mais reste exclusive de tout statut particulier. Nous devrons donc faire avec un « département doté de compétences différenciées », choix plus aisé, plaçant la collectivité alsacienne sur un chemin juridique balisé. Là encore, la jurisprudence constitutionnelle est aussi claire que bien établie : rien « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». Dans le cas qui nous occupe, chacun conviendra que, eu égard aux spécificités transfrontalières du territoire, nous nous inscrivons parfaitement dans un périmètre raisonnablement objectif pouvant appeler un traitement juridique particulier. Ainsi en est-il de ces avancées qui ont trait, entre autres, au plan sanitaire, au bilinguisme, mais aussi à la prise en compte, certes, de la de la situation très tendue du réseau routier national en Alsace du fait de l'existence de réseaux parallèles entre la France et l'Allemagne. Bien évidemment, nous savons que, pour l'essentiel, les compétences esquissées relèvent de logiques de planification, dont l'effet est nécessairement contraint. Cependant, il était important de fonder la particularité alsacienne autour d'un coeur de compétences confiées, à titre particulier à la Collectivité européenne d'Alsace, et d'asseoir ainsi la légitimité de l'évolution institutionnelle dans le passé tout autant que dans le futur. En tout état de cause, la voie de la collectivité à statut particulier, dont la fonction consiste à fonder son éloignement des cadres du droit commun, s'est malheureusement très vite heurtée à la vision d'un gouvernement soucieux de préserver l'édifice de la réforme régionale de 2015, qu'il n'entendait pas altérer. Ainsi, vous l'aurez compris, même si l'Alsacien que je suis aurait préféré aller plus loin et doter la collectivité de ce véritable statut particulier, je reconnais l'intérêt du compromis auquel nous sommes parvenus. Je tiens à le redire : le projet de loi que nous allons adopter aujourd'hui ne représente qu'une première étape de la démarche que nous avons engagée.

fort. Il fait partie d'un sujet plus large, celui de la décentralisation, répond à une demande réelle de la part des habitants et témoigne d'un engagement politique important des acteurs locaux relayé par les responsables nationaux.

L'Alsace est unique à bien des égards. Tout d'abord, son exception historique en fait un territoire clé, particulièrement sensible : en plus d'être le siège officiel du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, elle est une zone d'échange privilégiée. L'Alsace est dynamique sur le plan économique, avec deux aéroports et 62 000 travailleurs transfrontaliers. C'est un territoire agréable à vivre- réalité que l'on ne conçoit pas pleinement avant d'avoir entendu un Alsacien ou une Alsacienne parler de son territoire. Des cigognes sur les toits des églises, des maisons aux balcons fleuris, des forêts et même du vin : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, c'est un seul et même territoire avec une attractivité touristique exceptionnelle,

Le bilinguisme, la mobilité et le partage sont le résultat du caractère transfrontalier de ce territoire et de la recherche européenne de paix. L'Alsace est un exemple à suivre. On y vit pleinement et quotidiennement la citoyenneté européenne. Là-bas, nos voisins allemands sont dans tous les regards et à tous La création de la Collectivité européenne d'Alsace est en soi un nouvel acte de décentralisation, et le groupe Les Indépendants - République et Territoires s'en félicite ! Par ce projet de loi, le Gouvernement a pris en considération la spécificité de ce territoire, et c'est une réussite,

qui y vivent, là où ils savent qu'ils peuvent faire remonter les problèmes qu'ils rencontrent et les projets qui leur tiennent à coeur en s'adressant aux élus et aux acteurs locaux. Ce qui fait la richesse et la beauté de la France, c'est la diversité de ses territoires, de leurs paysages, de leurs spécificités. Ce qui est une réalité dans un territoire ne l'est pas forcément dans un autre. Les pouvoirs publics doivent s'adapter en fonction de cette diversité, la respecter et la valoriser. La décentralisation est avant tout une marque de respect envers la différence de ces territoires. Par la flexibilité qu'elle permet, elle est un élément décisif de la réussite économique. La cohésion territoriale passe par plus de souplesse, encourageant ainsi une dynamique de l'emploi et une concurrence saine. Elle favorise la vitalité des entreprises installées en province. Les décisions prises au plus près du terrain permettent une attention plus grande envers les différents acteurs. Ce projet de loi est un pas important dans la bonne direction ; il peut ouvrir la voie pour d'autres territoires. La Savoie, par

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je veux saluer le formidable travail accompli par toutes les parties prenantes. Ce projet de loi a été le fruit d'une initiative locale, notamment sous l'impulsion conjointe des exécutifs départementaux. Il a été Il a été discuté maintes fois avec le Gouvernement pour aboutir à la déclaration commune de Matignon, qui a servi de base politique sur laquelle les débats techniques ont pu s'engager. Nos débats se sont déroulés dans le respect de quelques grands principes. Tout d'abord, cette initiative législative est née, rappelons-le, d'une volonté alsacienne. En cela, elle ne devait reposer que sur le socle des intérêts alsaciens et il aurait été absolument infondé d'ouvrir une quelconque boîte de Pandore. pourquoi, dans un esprit de consensus, il n'appartenait pas au Sénat, représentant des collectivités territoriales, de s'opposer à une volonté locale sollicitant le concours du législateur. Ensuite, il était impératif de conforter la région Grand Est dans le champ de ses compétences, tout en honorant, dans un même geste, les engagements pris envers la Collectivité européenne d'Alsace nouvellement créée. Enfin, il revenait au processus parlementaire de s'emparer du débat autour de la différenciation territoriale et de parvenir à un point d'équilibre acceptable, tout particulièrement sur le calcul de la compensation du transfert des routes nationales, où, fort heureusement, le retour au droit commun s'est imposé. À l'issue de ce « numéro d'équilibrisme parlementaire », je crois également utile d'observer que ce texte de responsabilité et d'ouverture est d'abord le pari d'une méthode de bon sens, fondée sur la préfiguration législative, premier jalon de ce droit à la différenciation territoriale. En effet, ce texte nous offre en prime, à nous législateurs, une leçon d'humilité. Il nous rappelle qu'il ne peut y avoir un modèle d'organisation territoriale unique. De la même façon que l'on ne peut aplatir la réalité locale sous des considérations grossièrement universalistes, la décentralisation ne doit plus être un simple habillage, un prêt-à-porter. Elle exige des habits neufs, du « sur-mesure ». Notre groupe partage également une certaine idée de la République territoriale, fondée sur le cas par cas.

percevoir les enjeux par le prisme girondin ne suffira pas à renforcer notre République territoriale. De la même façon, la liberté locale ne se décrète pas à la faveur d'une révision constitutionnelle. C'est toute une révolution culturelle qu'il nous faut lancer. Mieux encore, c'est un élan de souplesse et un éloge de la diversité qu'il sera bon d'engager en faveur d'une société fondée sur la reconnaissance d'un droit à l'imagination créatrice des élus locaux. Aussi, le législateur ne doit pas perdre de vue que les lois de la République sont faites pour les citoyens, en l'occurrence, pour les Alsaciens et l'Alsace,

Je salue à cet égard le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, défendu par le ministre Sébastien Lecornu, qui partage cette logique de bon sens et dont le deuxième volet se traduira, dès le premier semestre de 2020, par la mise en oeuvre d'un acte de différenciation et de décentralisation. Ainsi, mes chers collègues, je témoigne ici de notre pleine adhésion au texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale n'aura pas mis fin à ce projet de création d'une Collectivité européenne d'Alsace. Elle l'aura à peine modifié. Pourtant, on ne pourra pas nous empêcher de penser que tout ce travail est brouillon et ne vise qu'à corriger les conséquences des dernières lois de réformes territoriales, voire à revenir en arrière sans avoir l'air d'y toucher. il est proposé de fusionner les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin afin de créer cette fameuse Communauté européenne d'Alsace, alors même que cette future structure recréera tout simplement la région Alsace démantelée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, et que la fusion des deux départements a été rejetée par référendum en 2013, avec un taux d'abstention record. Faut-il comprendre que la réforme des régions était une mauvaise loi ? Si l'Alsace renaît sous d'autres formes, pourquoi l'empêcherions-nous pour d'autres collectivités départementales ou régionales qui en feraient la demande ? Deuxièmement, il est transféré à cette nouvelle entité des compétences qui ne recouvrent ni totalement celles des régions ni celles des départements ! Ce texte crée donc bien un nouveau type de collectivité territoriale avec un droit dérogatoire- un super département au nom d'une différenciation territoriale qui n'est toujours pas inscrite dans notre Constitution et qui n'a donc aucune légitimité constitutionnelle. Si ! Là aussi, doit-on comprendre que la suppression de la clause de compétence générale des départements était une erreur que cette suppression ne permet plus l'expression des particularismes locaux ? Est-ce enfin la reconnaissance de l'échec de la loi NOTRe ? Apparemment non. On fera semblant de ne pas voir le problème global qu'entraîne ce texte, pour n'en corriger qu'à la marge les tares les plus flagrantes. on nous fait croire, avec ce texte, qu'en l'état actuel il serait impossible à ces départements de mettre en place des politiques de coopérations transfrontalières. C'est tout simplement faux Les collectivités frontalières n'ont pas attendu ce texte pour s'atteler à ce sujet. Consacrer de cette manière la volonté de réduire les frontières en ouvrant la voie à une telle zone franche franco-allemande peut en revanche inquiéter quant à l'alignement par le bas, le fameux dumping social, mais aussi environnemental, du fait de l'explosion du transport routier qui pourrait advenir au nom

continuent de penser, comme l'a rappelé Pierre-Yves Collombat lors de la première lecture au Sénat que « le jacobinisme français- comme certains le dénomment -n'est pas qu'un centralisme : c'est un étrange mélange de centralisme et de liberté locale » et « dans le système administratif classique, le préfet et son administration ne sont pas que la courroie de transmission de l'État central ; ils sont aussi les porte-parole des territoires et de leurs élus auprès de l'État ». En clair, le triptyque communes-départements-État, issu de la Révolution française, reste un outil d'une grande efficacité et d'une grande souplesse, qui a permis unité et prise en compte des particularismes, sans mettre en concurrence les territoires. C'est pourquoi nous ne saurions soutenir un texte qui, peut-être sans s'en rendre compte, favorise un projet institutionnel libéral, qui passe par la création d'un nouveau triptyque EPCI-régions-Europe, qui signerait, en l'affaiblissant, la fin de la légitimité de l'État-nation. Voilà pour la vision globale que le groupe CRCE porte sur ce texte. J'en viens à ses détails. L'article 2 donne compétence à cette nouvelle entité en matière de tourisme et de promotion de l'attractivité du territoire, tout en s'assurant que l'exercice de cette compétence reste compatible avec les schémas régionaux.

Encore une fois, quelle est la logique, si ce n'est un désengagement à pas feutrés de l'État dans les territoires ? à la différence territoriale, ce bricolage législatif, ni fait ni à faire, est une nouvelle étape de l'opération de démembrement de la République indivisible qui porte le nom de France. C'est pourquoi le groupe CRCE ne votera pas ce texte, prélude à une inégalité accrue des territoires.

lorsqu'ils font visiter ce magnifique édifice de la République qu'était le palais de Marie de Médicis, les guides rappellent

dans l'esprit du droit à la différenciation annoncée par le Président de la République, qui ne voit pas encore le jour, puisque la réforme constitutionnelle ne se fait pas -quelques compétences spécifiques. Dans ces

Nous l'avions fait à propos de la coopération transfrontalière, en allant un peu plus loin que ce qui se fait aujourd'hui et en essayant de voir comment l'État, qui est loin d'être facile, pouvait donner à des collectivités frontalières des compétences déléguées pour agir.

Autre domaine de compétence, le bilinguisme. Je reprends à mon compte les propos de notre collègue Guy-Dominique Kennel, qui était à l'époque président du conseil départemental du Bas-Rhin et qui sait parfaitement que le bilinguisme et la convention qui est visée dans ce texte existaient déjà.

c'est totalement impossible. Cela rassurera nos amis lorrains, qui avaient obtenu du Sénat, à l'unanimité des présents, y compris des Alsaciens, que ce qui se fera pour l'A35 puisse se faire aussi pour les routes de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

depuis plusieurs années, les départements sont présentés comme ayant vocation à s'effacer, absorbés ici par les régions, happés là par les métropoles. Au fil des lois, des éléments devant conduire à " constater leur inutilité " sont distillés, comme le préconisait le rapport Attali de 2008, inscrivant cet objectif dans un délai de dix ans. Et pourtant, force est de constater que les départements sont toujours présents, paraissant même ragaillardis par les batailles qu'ils livrent, mais peut-être contraints de se découvrir quelque peu autres Ainsi s'exprimait fort justement Nelly Ferreira, professeure de droit public, dans un récent article illustrant parfaitement la situation en Alsace. À l'inverse de leur disparition est créé est créé un nouveau grand département d'Alsace- il s'agit bien d'un département, comme l'a rappelé le Conseil d'État -, appelé Collectivité européenne d'Alsace, réunissant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais doté de compétences supplémentaires, notamment étatiques. Si nous comprenons bien qu'un « désir d'Alsace » ait pu émerger pour des raisons historiques et qu'il se soit érigé ensuite dans une posture défensive par rapport à la région Grand Est, notre devoir de parlementaire est d'examiner le projet de loi à l'aune du caractère indivisible de notre République et du principe d'égalité entre tous les citoyens. « Du cousu main » : ainsi était qualifié l'accord de Matignon pour la création d'une Collectivité européenne d'Alsace. nous nous interrogeons sur la rigueur de la méthode : pourquoi se réduire à compenser les erreurs originelles de la loi Maptam et de la loi NOTRe au cas par cas, en fonction des mécontentements ? Les débats au Sénat ont conduit à l'adoption, à l'article 1, de l'amendement de notre collègue François Grosdidier généralisant à tous les départements qui en feraient la demande les compétences attribuées à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace- cette disposition a été supprimée par la suite en commission mixte paritaire. Pour des raisons de cohérence, nous étions opposés à cet amendement traitant des compétences de l'ensemble des départements dans une loi traitant spécifiquement de la Collectivité européenne d'Alsace et nous étions contre l'idée de revenir à une France « cousue main » d'avant la Révolution.

Il a également été soutenu que cette nouvelle entité serait un prélude à un mouvement plus large fondé sur le futur droit à la différenciation. Nous aimerions que cet accord, qui procède strictement d'un tête-à-tête entre deux départements, une région et l'État, ne vienne pas préfigurer le futur droit à la différenciation, sur lequel les parlementaires doivent encore s'accorder entièrement. La différenciation reste un risque pour l'égalité territoriale. Il faut pouvoir l'accompagner de garde-fous et le débat parlementaire doit bien entendu trouver un juste équilibre. L'examen que nous avons fait de ce texte sur l'Alsace, circonscrit uniquement à des séances publiques de nuit, aussi riches que les débats aient été, ne saurait en aucun cas préfigurer une réforme si complexe. en outre quelques réserves du point de vue de l'organisation territoriale et administrative telle qu'elle est prévue dans le texte. Nous continuons à nous interroger sur la création de doublons- d'État avait relevé ce point -, avec le maintien des deux circonscriptions administratives et des préfectures de Colmar et de Strasbourg en parallèle du nouveau département d'Alsace. Enfin, à l'image de cette nouvelle Collectivité européenne d'Alsace, mais aussi des intercommunalités « XXL » ou des grandes régions, les autres départements ont-ils vocation à se livrer à des jeux de fusion pour pouvoir continuer à développer leurs projets et servir de refuge entre deux réformes structurelles ? Il existe peut-être une alternative permettant aux territoires de mener correctement leurs projets : retrouver le sens de la libre administration, laisser les collectivités décider dans leurs domaines de compétence et mettre un frein à l'inflation normative et législative.

Un grand nombre de collègues du RDSE reste sceptique sur le présent projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace pour trois raisons principales : il ouvre la voie à une organisation territoriale à géométrie variable, que nous réfutons nous contestons la méthode avec laquelle la question de la différenciation territoriale est amenée ; nous estimons que la loi n'a pas à arbitrer un par un tous les cas particuliers. apportera en revanche sa contribution au nouvel acte de décentralisation et estime que celui-ci aurait dû constituer le cadre d'une telle évolution. Mes chers

l'alimentation. Monsieur le ministre, après l'épisode de l'an dernier, la France connaît de nouveau une grave sécheresse et les canicules à répétition n'arrangent rien. Cette sécheresse touche la métropole, mais aussi les outre-mer, comme l'île de la Réunion ou celle de la Martinique. Le monde agricole est l'une des premières victimes de ces événements. Certes, vous avez déjà annoncé quelques mesures. Comme l'an dernier, le dispositif de calamité agricole sera activé, les constructions de retenues collectives d'eau de pluie sont autorisées depuis le mois dernier et des flux de solidarité entre des départements disposant de fourrage et ceux qui en manquent seront mis en place. Vous allez solliciter de l'Union européenne le déblocage en octobre de 70 %, au lieu de 50 %, des aides de la politique agricole commune, mais cette avance de trésorerie n'arrivera qu'après la sécheresse, c'est-à-dire trop tard Nous ne pouvons pas accepter que nos éleveurs doivent se résigner à envoyer leurs bêtes à l'abattoir, parce qu'ils n'ont plus de quoi les nourrir. Nous devons trouver des solutions pour la sécheresse de cette année, mais aussi pour celles qui suivront. La France doit se préparer à subir régulièrement de tels épisodes. La réponse de l'État doit être anticipée. Monsieur le ministre, pouvez-vous faire un point sur la situation actuelle et nous dire quelles mesures vous envisagez à court et moyen terme ? La parole

pour autoriser la construction de retenues d'eau à multi-usages, qui doivent permettre l'irrigation de l'agriculture. C'est très important ! Le problème auquel nous sommes confrontés- je livre ce constat à la Haute Assemblée qui est une assemblée de sages -, c'est qu'avant même la mise en place d'un projet

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Dans un État de droit, il revient à l'État d'assurer le respect des lois de la République et la sécurité de chacun de nos concitoyens sur tout le territoire national, en tout temps et en toutes circonstances. Après près de neuf mois où le rendez-vous hebdomadaire des Français était le journal de 20 heures du samedi soir pour connaître l'étendue des dégâts occasionnés par les « gilets jaunes », certains ont vite compris qu'ils pouvaient insulter, casser, piller, profaner, voire agresser dans la plus totale impunité. Ainsi, dans mon département du Val-de-Marne, à peine installés, les mâts des caméras de vidéosurveillance ont été sciés à la meuleuse par les dealeurs à Villejuif et dans plusieurs autres communes. La ville de Limeil-Brévannes connaît, elle, des actes d'une violence inédite : quinze véhicules ont été incendiés devant la mairie ; l'hôtel de ville et le centre socioculturel ont été attaqués à la voiture bélier enflammée, en représailles à l'arrestation de quelques trafiquants qui s'en vantent.

Il n'est pas acceptable que, dans notre démocratie, des voyous attaquent et détruisent les symboles de la République, persuadés, s'ils sont identifiés, de s'en sortir avec une simple relaxe. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour rétablir l'ordre républicain dans nos territoires, notamment aujourd'hui à Limeil-Brévannes

J'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec Mme la maire de cette commune et elle a été reçue hier par mon cabinet avec le député Laurent Saint-Martin pour trouver les moyens de faire face à cette situation. Que s'est-il passé précisément dans cette commune ? Il se trouve que, le 1 juillet, nous avons démantelé un important réseau de trafic de drogue, nous avons saisi 100 000 euros et interpellé sept personnes qui ont été placées sous écrou. Et nous subissons la réaction de ces voyous et de leurs amis.

un plan d'action qui refonde en profondeur la lutte contre les produits stupéfiants sur l'ensemble du territoire ; nous le présenterons à la rentrée avec des moyens nouveaux. Aucun mètre carré

dans mon département, le Loir-et-Cher, l'un des départements français les plus touchés par l'épisode de sécheresse qui frappe la France depuis plusieurs semaines et qui touche tous nos compatriotes. Je tiens à souligner votre engagement auprès de nos agriculteurs. Ainsi, vous avez annoncé le versement anticipé d'une partie des aides européennes dédiées à l'agriculture, ainsi que l'autorisation donnée aux éleveurs de faucher les jachères pour nourrir le bétail. Ces annonces vont dans le bon sens, mais elles constituent des réponses de court terme pour parer à l'urgence. Le dérèglement climatique fait craindre des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Il nous faut donc mettre en place des outils durables pour protéger les agriculteurs français et préserver notre modèle agricole. Nous devons revoir en profondeur notre approche et nos méthodes agricoles. Cela commence par un travail sur le stockage de l'eau et le développement de l'irrigation. Nos agriculteurs font des efforts très importants pour utiliser moins d'eau et irriguer toujours plus efficacement. Cependant, tant que la France n'adoptera pas des méthodes de captation de l'eau beaucoup plus efficaces, nous ne pourrons pas anticiper et lutter contre la sécheresse. Sur ce point, l'État a un rôle majeur à jouer, notamment en simplifiant les procédures administratives pour la création des retenues collinaires. Monsieur le ministre, je vous sais impliqué sur ce sujet qui a été abordé lors des dernières assises de l'eau. La vague actuelle de sécheresse le montre : il faut aller plus vite et plus loin. Les professionnels du monde agricole sont disposés à avancer avec vous sur ce point majeur. Il faut fixer un calendrier précis, des objectifs concrets et lever les barrières administratives qui empêchent notre agriculture de se transformer aussi vite que le climat. Monsieur le ministre, pouvez-vous détailler les mesures qui seront prises par le Gouvernement pour répondre rapidement et efficacement à la question majeure du stockage et de l'utilisation de l'eau dans le secteur agricole ? Merci d'avance

pour obtenir la possibilité de faucher des jachères dans 24 départements plus 9, soit 33. Ce n'est pas assez et je veux continuer la bataille dans les jours qui viennent pour que la Commission européenne ouvre les yeux et se rende compte que la sécheresse est forte dans de très nombreux départements. Nous devons aller plus loin et pouvoir faucher les jachères dans d'autres départements afin de donner à manger au bétail et éviter les difficultés que nous avons connues l'année dernière. De plus, il faut absolument que nous obtenions de la Commission

Le troisième point, c'est de demander à l'ensemble des agriculteurs qu'ils ne broient plus les pailles pour la méthanisation. L'heure est grave, il faut tout mettre sur la table pour que la solidarité joue à plein. Or les agriculteurs sont des gens qui savent ce qu'est la solidarité.

À la suite de l'incendie du CHU de Guadeloupe le 28 novembre 2017, tous les services connaissent une désorganisation, en particulier les urgences et les trois unités de médecine néonatale. Madame la ministre, nous connaissons votre implication sans cesse manifestée auprès de nos professionnels de santé. la situation catastrophique, maintes fois signalée par les agents et les médecins, n'a, jusqu'à ce jour, pas reçu de réponse satisfaisante à la hauteur des enjeux sanitaires. Au moment où je vous parle, le personnel est en grève. Vous comprendrez aisément le ras-le-bol des professionnels de santé, qui, tous les jours, font des prouesses pour maintenir la sécurité et la continuité des soins. À toutes ces difficultés s'ajoute la situation très largement dégradée des finances de l'établissement, qui ne peut assurer dans de bonnes conditions l'approvisionnement des denrées et des médicaments pour les patients. Les parlementaires, notamment le député de la circonscription, Olivier Serva, l'ont déjà signalé. Pour rappel, à ce jour, la dette du CHU envers ses fournisseurs avoisine les 49 millions d'euros.

Madame la ministre, les attentes sont fortes et la détermination professionnelle des agents est encore intacte. Ces derniers attendent, au-delà des discours rassurants, des signaux tangibles, un vrai plan Marshall, mais également une déclinaison de la stratégie de reconquête de la population envers son CHU. La prévision d'ouverture du nouvel établissement dans les cinq prochaines années ne doit en aucune manière occulter la nécessité du maintien du niveau de soins des patients. Cette évidence conduit d'ores et déjà la collectivité régionale à soutenir, au côté de l'État, le projet d'équipement d'une salle de coronarographie interventionnelle, investissement ô combien important pour la bonne prise en charge de nos patients. Pourriez-vous, madame la ministre,

Théophile, le CHU de la Guadeloupe occupe effectivement une place prépondérante dans l'offre de soins de ce territoire et je suis extrêmement vigilante, depuis cet incendie, à ce que cet établissement soit capable de remplir les missions qui sont les siennes envers la population guadeloupéenne. La situation particulière relative au paiement des fournisseurs, que vous citez, est suivie attentivement par l'agence régionale de santé et par mon ministère. Un plan d'apurement de la dette a été établi et une aide supplémentaire en trésorerie a été versée à l'établissement début juillet, laquelle permettra d'atteindre, au total, 48 millions d'euros d'aide pour pour les six premiers mois de 2019, ce qui devrait permettre d'accompagner la résorption progressive de la dette. Une ligne de secours en trésorerie a également été mise en place, conformément au souhait du Président de la République, sous la forme d'un « bon à tirer » par le directeur de l'établissement en cas de nécessité ou d'urgence. Je tiens à saluer l'engagement des équipes du CHU qui effectuent, vous avez raison de le rappeler, un travail absolument remarquable pour prendre en charge les patients dans des conditions que je sais difficiles en raison de la dispersion des sites sur l'île. Le plan de réorganisation de l'offre de soins est suivi et la situation structurelle de l'établissement devrait être stabilisée, comme prévu, en 2020. Ce plan a fait l'objet d'un financement important, à hauteur de 54 millions d'euros, pour la livraison d'un nouveau pôle parents-enfants en octobre 2020 pour la réhabilitation des premiers services, dont les urgences, d'ici à la fin de l'année. Les blocs seront de nouveau opérationnels au premier semestre 2020. Enfin, nous resterons tous mobilisés pour que la construction du nouveau CHU se fasse le plus rapidement possible je renouvelle ma confiance à la directrice de l'ARS comme au directeur général du CHU pour mener à bien ces actions et cette réorganisation. Je remercie également la collectivité régionale de son aide, laquelle est déterminante pour que ces réorganisations soient cohérentes avec les besoins de santé du territoire. La parole

C'est pour cela que nous défendons ceux qui se sentent parfois oubliés par Paris et qui subissent à la fois le recul des services publics et les effets délétères de l'enclavement. Je ne vous apprends pas que l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 kilomètres à l'heure sur certaines routes a été vécu par beaucoup comme une mesure vexatoire, totalement déconnectée des réalités. En réaction, le Sénat, dans sa grande sagesse, a voté le 20 février dernier, sur notre initiative, la possibilité de relever à 90 kilomètres à l'heure la limitation de vitesse sur certaines routes départementales et nationales. La LOM, qui sera examinée en nouvelle lecture à la rentrée, a introduit un dispositif de même nature. La cause semblait donc entendue. Pourtant, le Conseil national de la sécurité routière a publié la semaine dernière une grille d'analyse, c'est-à-dire une série de six recommandations destinées à « accompagner les décisions des élus », parmi lesquelles : « énoncer l'objectif recherché et les gains à retirer d'un relèvement de la vitesse », ou identifier des tronçons homogènes d'une longueur minimale de 10 kilomètres sans traversée d'agglomération. Au-delà de ce vocable administratif, beaucoup de conseils départementaux s'interrogent aujourd'hui sur la valeur à accorder à ces recommandations, craignant surtout que l'on ne leur retire d'un côté la latitude d'action qu'on leur a rendue de l'autre. Monsieur le Premier ministre, personne ici ne contestera la nécessité de faire mieux en matière de sécurité routière, mais personne ne veut non plus qu'il subsiste des citoyens de seconde zone. Pouvez-vous alors nous éclairer sur le statut de ces recommandations et, surtout, rassurer l'ensemble des élus locaux, eux qui connaissent le mieux nos territoires ? Bravo, il a raison ! La parole est à M. le Premier ministre.

dans le cadre des comités départementaux de la sécurité routière. Elle leur permettra de choisir la façon dont ils veulent organiser les choses sur ce réseau. Il ne s'agit pas de revenir en quoi que ce soit sur cette possibilité offerte aux présidents de conseils départementaux, dont certains ont indiqué qu'ils voudraient se saisir quand d'autres, d'ailleurs, ont affirmé qu'ils ne souhaitaient pas changer la limitation à 80 kilomètres-heure.

s'agit d'un de ces organismes composés d'experts, d'élus locaux et nationaux. Il a formulé des aides à la décision, des recommandations,

Cette recommandation me paraît empreinte de bon sens et d'expertise, mais il appartiendra, bien entendu, à ceux qui sont les gestionnaires des réseaux de prendre leurs responsabilités ; c'est tout le sens de la LOM ; c'est tout le sens de la LOM et de ce que nous avons voulu mettre en oeuvre. Pour sa part, l'État, qui est lui aussi gestionnaire d'une partie du réseau concerné, a fait le choix de fixer la la limitation maximale à 80 kilomètres-heure, un choix qu'il assume par la voix du Premier ministre, chef du Gouvernement. Il appartiendra aux présidents des conseils départementaux d'utiliser la faculté qui leur sera ouverte par la loi d'orientation sur les mobilités, lorsqu'elle aura été publiée,

la direction de Conforama veut licencier 1 900 salariés et fermer 32 magasins. Elle les liquide, au coeur de l'été, comme d'autres abandonnent leurs chiens sur le bord de la route des vacances. Conforama, c'est l'histoire trop banale du capitalisme mondialisé : un groupe qui n'investit plus et se contente de gérer une rente ; un investisseur étranger, déguisé en chevalier blanc, qui falsifie ses comptes pour fondre sur une proie juteuse l'État français qui lui accorde, en guise d'absolution, des avantages fiscaux à hauteur de 63 millions d'euros ; enfin, une reprise qui tourne au fiasco et menace 9 000 salariés. Comme toujours, les actionnaires du groupe prédateur, Steinhoff, en l'occurrence, ont déjà sauvé leur mise en vendant tout ce qui pouvait l'être. La semaine dernière, dans ce même hémicycle, vous aviez pris, madame la secrétaire d'État, l'engagement d'une action ferme pour obtenir de la direction de Conforama des garanties sur la pérennité du groupe et sur la sauvegarde de l'emploi. Où en êtes-vous ? Sur le fond, alors que votre gouvernement ne cesse de dénoncer l'addiction à l'argent public, quand allez-vous soumettre l'octroi d'aides de l'État au respect d'engagements en faveur de l'emploi, de l'investissement et des droits sociaux ?

tant à l'actionnaire qu'à l'ensemble de l'entreprise. Ces efforts se poursuivent aujourd'hui. Au-delà des difficultés de son actionnaire, le groupe Conforama doit faire face, comme beaucoup d'acteurs de la distribution, à une transformation majeure des modes de consommation à la concurrence croissante des acteurs de l'économie numérique. Vous le savez, Conforama perd beaucoup d'argent, mais aussi des clients. Pour faire face à ces défis, le groupe doit maintenant se transformer afin de répondre

la fermeture de 32 magasins et de 10 magasins Maison Dépôt. Après l'émotion importante et légitime qui s'est manifestée lors de l'annonce de la restructuration, les négociations autour du plan social se sont engagées. Notre souhait est que la direction et les organisations syndicales poursuivent ce dialogue de manière transparente et loyale. Le Gouvernement a pour objectif d'assurer la pérennité de ce groupe, qui compte près de 9 000 emplois en France. Nous serons donc particulièrement attentifs quant aux conditions de mise en oeuvre de la restructuration, doit donner à l'entreprise toutes ses chances de poursuivre son activité. Mes services et moi-même serons également particulièrement vigilants quant aux efforts de reclassement et aux mesures d'accompagnement qui seront mises en place par le groupe. C'est maintenant que la négociation commence. La parole

Par ailleurs, les ménages, qui contribuent à 60 % aux prélèvements obligatoires, auront une nouvelle fois le sentiment que leurs impôts récompensent des entreprises qui se servent et qui privilégient leurs intérêts financiers à court terme.

la chronique alors qu'il envisageait la reprise d'Ascoval, vient d'être placé en redressement judiciaire. Il a également annoncé mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour sa filiale implantée à Cosne-sur-Loire et à Tarbes, avec un risque de fermeture définitive des deux sites. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma solidarité à l'égard des salariés de l'entreprise, qui vivent une situation inconfortable depuis 2016. Il faut savoir qu'alors votre prédécesseur, M. Macron, s'était engagé dans cet hémicycle à recapitaliser le groupe Vallourec en contrepartie de restructurations limitées et de la réalisation d'investissements sur les sites concernés. Deux ans après ces annonces, l'entreprise Vallourec a cédé ces sites à Altifort, qui s'était alors engagé à conserver les effectifs pendant au moins deux ans. Aujourd'hui, on sait que cet engagement ne sera pas tenu ! Devant cette situation, nous ne pouvons que relever une quadruple responsabilité : celle de Vallourec, dont l'État est le principal actionnaire et qui a choisi le groupe Altifort parmi les repreneurs potentiels ; celle de la société d'accompagnement à la reprise, dont les analyses ont servi à qualifier Altifort ; celle d'Altifort et de ses dirigeants, qui n'ont pas utilisé la totalité des 10 millions d'euros que Vallourec leur avait alloués pour relancer le site, puisque 3 millions d'euros ont été transférés à la holding dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie et font aujourd'hui défaut dans les caisses de la filiale cosnoise ; celle, enfin, de l'État, qui, dès le début de l'opération, a apporté sa caution. Alors que le Président de la République a annoncé l'ouverture d'une usine Safran près de Lyon avec 250 emplois à la clé, quelle est la politique industrielle de l'État à destination des territoires non métropolitains qui ont une histoire et une actualité industrielles et qui souhaitent avoir un

et ses deux sites de Tarbes- 45 salariés -et de Cosne-sur-Loire- 117 salariés. Vallourec a cédé l'activité Drillà l'Américain NOV fin 2017 ; je rappelle que cette cession s'est faite dans de très bonnes conditions et que les salariés repris

mentionnez se fasse dans les meilleures conditions et que l'on assure le rebond de ces salariés dans une zone où l'on doit pouvoir retrouver de l'emploi industriel. Aujourd'hui, en effet, 50 000 emplois industriels sont à pourvoir.

pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Au mois de juillet 2017, vous assuriez, monsieur le Premier ministre, dans votre discours de politique générale, que le Gouvernement tiendrait la promesse du candidat Emmanuel Macron de créer 15 000 places supplémentaires de prison.

Or il semble aujourd'hui que ce chiffre ne sera pas atteint. En effet, dans le rapport au Parlement sur l'orientation budgétaire, le Gouvernement vient d'annoncer la révision à la baisse des crédits du ministère de la justice, remettant ainsi en cause la trajectoire adoptée il y a cinq mois à peine et que le Sénat avait déjà jugée insuffisante. Par rapport aux engagements votés dans la loi de programmation, on peut craindre un différentiel de 200 millions d'euros. Rapporteur de la mission « Justice », je suis particulièrement inquiet de cette baisse envisagée des crédits, qui ne peut qu'emporter des conséquences désastreuses sur une situation carcérale déjà fortement dégradée comme sur le fonctionnement général de nos juridictions. Aussi, monsieur le Premier ministre, ma question est simple : pouvez-vous nous rassurer sur les moyens attribués au ministère de la justice afin, en particulier, de tenir au moins l'objectif des 7 000 places de prisons annoncées et de permettre à notre justice d'avoir des moyens dignes d'une démocratie du XXI siècle ? La parole

la question. Je tiens à réaffirmer devant vous que nous livrerons en 2022 la plupart des établissements qui ont été promis et que nous poserons les premières pierres des établissements prévus

Enfin, s'agissant des prisons, nous savons que les conditions actuelles de détention ne permettent ni leur bonne gestion, ni la réinsertion de nos détenus, ni une lutte efficace contre la radicalisation et contre les différentes formes de violences. Avec mes collègues des commissions des finances et des lois, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine discussion du budget de la mission « Justice », au cours de laquelle chacun devra prendre ses responsabilités.

Cartron, pour le groupe La République En Marche. Ma question s'adresse à Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Depuis deux ans, l'orientation des étudiantes et des étudiants dans l'enseignement supérieur public s'effectue au travers du système Parcoursup.

La phase principale d'admission dans l'enseignement supérieur s'est achevée jeudi dernier, conformément au calendrier accéléré que vous nous aviez annoncé ici même. Neuf bacheliers sur dix ont d'ores et déjà reçu une proposition d'admission. nombreuses réussites et à eux aussi de bonnes vacances ! Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que Parcoursup a encore mieux fonctionné en 2019 que l'année précédente et qu'il répond toujours mieux aux exigences de mixité sociale dans les filières du supérieur ? Nous pensons également aux étudiants qui n'ont toujours pas reçu d'affectation à ce jour, alors que la phase complémentaire se poursuit jusqu'au 14 septembre et qu'un peu plus de 90 000 places sont toujours disponibles. Quels dispositifs d'accompagnement et d'aide leur sont proposés afin que leur recherche aboutisse le plus rapidement et le mieux possible ? Merci de votre écoute

oui ! ... le logiciel qui permet l'orientation des étudiants est venu en remplacement d'admission post-bac, lequel, je vous le rappelle, tirait au sort nos jeunes pour leur faire intégrer l'enseignement supérieur. Parcoursup, en tant que logiciel d'orientation, s'appuie aussi sur une confiance renouvelée à la fois dans les professeurs du secondaire et dans les professeurs du supérieur, qui, au côté des conseillers d'orientation, permettent d'améliorer les choix faits par les étudiants et leurs familles.

l'équité et la justice. Depuis 2008, une convention exige que l'Unédic verse 10 % des cotisations chômage collectées pour assurer le fonctionnement de Pôle emploi.

On comprend d'autant moins cette ponction que certains sont dispensés de l'effort commun. En effet, le Gouvernement a décidé de ne demander aucun effort aux intermittents du spectacle, qui ne seront pas concernés par la réforme de l'assurance chômage. pourtant, l'indemnisation et l'accompagnement dans l'emploi de 120 000 intermittents ont coûté 1,3 milliard d'euros, pour seulement 367 millions d'euros de recettes, soit un déficit de 1 milliard d'euros. Les intermittents sont donc largement bénéficiaires de l'assurance chômage. Madame la ministre, après la colère des « gilets jaunes », les Français demandent que les réformes soient équitables et mises en oeuvre dans un esprit de justice. Tout le monde devrait donc contribuer à la réforme ! Ce sont les salariés, la CSG et les cotisations chômage, qui financent majoritairement le fonctionnement du service public de l'emploi. Pour quelles raisons les intermittents du spectacle restent-ils intouchables et épargnés par cette réforme ?

inciter au retour à l'emploi les demandeurs d'emploi ; mieux accompagner ces derniers, pour que le retour à l'emploi soit plus rapide et plus efficace. Le passage de 10 % à 11 % de la cotisation permettra ce renforcement inégalé

des salariés du secteur du spectacle. La nouvelle convention des intermittents du spectacle, qui date de 2016, doit maintenant être évaluée. Il n'y a pas lieu, pour l'instant, de changer ce régime, qui obéit déjà à des conditions très particulières. Vous verrez,

le texte était voté, douze jours plus tard, dans notre assemblée. Depuis lors, nous pouvons considérer que, quelle que soit la nature du crime commis en France, la justice rendue au nom du peuple français ne s'abaisse plus à la barbarie en prononçant la peine capitale. La France n'a jamais cessé de réaffirmer dans le cadre des Nations unies, à l'assemblée générale comme au conseil des droits de l'homme, son attachement à l'abolition de la peine de mort dans le monde et soutenu à de nombreuses reprises des résolutions à visée abolitionniste. Néanmoins, un certain nombre de nos compatriotes se trouvent aujourd'hui sous le coup d'une condamnation à mort, dans des pays où cette peine n'a pas encore fait l'objet d'une abolition. Le dernier d'entre eux, un Béthunois de 35 ans, a été condamné à la peine capitale par un tribunal indonésien, le 20 mai dernier, rejoignant ainsi la triste liste des ressortissants français

Sans remettre en cause la souveraineté judiciaire de ces États, la France, qui a inscrit l'interdiction de la peine de mort dans sa Constitution, ne peut rester inerte quant à l'intégrité physique de ses ressortissants

apporter soutien et information à leur famille

vous l'avez souligné, la France rappelle en permanence son opposition totale à la peine de mort, quels que soient les crimes, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances. Ce combat en faveur de l'abolition universelle constitue l'un des axes forts de notre diplomatie, qui agit au sein des enceintes multilatérales, mais aussi des pays non abolitionnistes, pour que ce principe fondamental de la manière de vivre ensemble, si je puis dire, soit adopté par l'ensemble des pays. Nous essayons aussi, dans la mesure du possible, d'agir auprès des pays directement concernés que je viens de citer, pour que les autorités puissent commuer la peine de mort en une autre peine.

ce qui se traduit par un contact régulier avec notre poste consulaire, des visites régulières sur son lieu de détention, un accompagnement de sa famille et un accompagnement auprès des autorités indonésiennes. Là comme ailleurs,

de développer leur sens critique, d'évaluer celles et ceux qu'ils ont élus pour les représenter. Or il est malheureusement évident que les entraves à la liberté d'expression se multiplient dans notre pays la transposition de la directive européenne sur les affaires, qui vise à protéger nos secrets industriels, permet à des grands groupes de faire taire la presse ; la loi contre les fausses informations pourra également s'appliquer aux informations qui ne peuvent être vérifiées, avec un risque de retour à la censure la loi contre la haine sur internet permettra à des hébergeurs ou, pis, à des algorithmes de s'ériger en censeurs et de supprimer arbitrairement certains contenus. s'ajoutent les déclarations, puis le rétropédalage du Gouvernement sur la création d'un conseil de l'ordre des journalistes. Sans parler des journalistes sommés de dévoiler leurs sources aux services de renseignement dans le cadre, par exemple, des Yémen Papers et de l'affaire Benalla. Ces textes Ces textes de loi répondent, certes, à de vraies problématiques, mais, mal utilisés ou détournés, ils représentent un vrai danger pour les libertés publiques. Que comptez-vous faire pour sanctuariser la liberté de la presse ?

nationale. Je partage évidemment avec vous la conviction que l'État doit être le garant des libertés publiques, parmi lesquelles figure, sans doute au premier rang, la liberté d'information. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait de cette liberté un principe fondamental, « un des « un des droits les plus précieux de l'homme ». Cette liberté a évidemment pour corollaire le fait de protéger en tout temps et en tout lieu la profession de journaliste, dont l'exercice libre est indispensable à celui de notre démocratie L'exercice de la profession de journaliste est fondé, vous l'avez rappelé, sur le principe de la protection des sources. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même fait de la protection des sources une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Notre législation s'y attache également, au travers de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, aux termes de laquelle il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. C'est avec cette conviction que le Premier ministre a échangé avec un certain nombre de professionnels. Le Gouvernement avait confié à M. Emmanuel réflexion sur la mise en place d'un conseil de déontologie des médias, qui serait une forme d'instance d'autorégulation de la profession. Cette question peut être légitimement posée, au vu de l'évolution de la profession et du développement des réseaux sociaux. Une telle instance existe d'ailleurs chez un certain nombre de nos voisins.

madame la secrétaire d'État, il ne suffit pas de dire que la liberté de la presse est et sera toujours respectée pour que le but soit atteint.

Sous couvert de sécurité nationale, de secret des affaires, de lutte contre les ou contre la haine sur internet, ne construisons pas, brique par brique, le mur de la désinformation

La séance est reprise. Nous reprenons l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la bonne politique, c'est l'art du possible la récente histoire institutionnelle de l'Alsace en est un bel exemple. L'Alsace n'a pas de problème d'identité dans les coeurs et dans les esprits. Son problème, depuis son incorporation dans la région Grand Est, c'est d'exister de nouveau dans les institutions de la République.

je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration et au vote de ce texte. Je tiens à mentionner plus particulièrement Mme Jacqueline Gourault, qui a conduit la concertation, le président de notre commission des lois, M. Philippe Bas, et la rapporteur du projet de loi, Mme Agnès Canayer, qui se sont pleinement investis pour permettre la concrétisation du « désir d'Alsace ». À titre personnel, en tant qu'initiateur de l'amendement qui a permis le rétablissement de la dénomination « Collectivité européenne d'Alsace »,

La loi sera complétée par différentes mesures qui relèvent du pouvoir réglementaire de l'État. En particulier, le retour des statistiques à l'échelle de l'Alsace et des plaques minéralogiques alsaciennes aura une portée politique évidente.

collectivité. Ce qui compte en politique, c'est la perception que l'on a d'un événement. À cet égard, la Collectivité européenne d'Alsace a été accueillie avec une satisfaction profonde par les deux conseils départementaux, qui en avaient approuvé le principe à la quasi-unanimité-

Quant aux régionalistes autonomisants, ils déplorent que l'Alsace, à défaut de sortir du Grand Est, n'ait pas obtenu le statut particulier qu'ont la Corse, Paris et Lyon. Je rappelle que le statut particulier de ces collectivités résulte de la fusion de deux assemblées de nature différente. Ce statut, les Alsaciens l'ont laissé passer avec le référendum raté de 2013 sur la fusion des deux conseils généraux et du conseil régional. Je suis d'un naturel optimiste et réaliste, ce qui m'a permis d'être élu local, régional, puis national depuis quarante-huit ans. Je vois donc naturellement le verre à moitié plein Certes, je n'ignore pas les points d'insatisfaction de ce projet de loi, mais nous avons abouti à une rédaction qui va, pour l'essentiel, aussi loin que possible dans le cadre constitutionnel existant, sans enclencher le détricotage de la carte des régions de France. La révision de la Constitution ouvrira également de nouvelles perspectives à l'Alsace, avec le droit à la différenciation. Finalement, cette loi constitue une avancée par rapport à la situation existante depuis 2014, et si la Collectivité européenne d'Alsace fait preuve de son efficacité dès le 1 janvier 2021, ce dont je ne doute pas, rien

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au bout du parcours parlementaire sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace,

À la première question, je ne suis pas certain que l'on puisse répondre par l'affirmative. En matière de renforcement du bilinguisme comme de soutien aux activités du territoire, l'écriture du projet de loi s'éloigne singulièrement du texte de la déclaration. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre sur ce point,

Enfin, pour l'anecdote, si conformément à la déclaration de Matignon, les fédérations culturelles et sportives peuvent organiser leur gouvernance infrarégionale à l'échelle alsacienne, elles ne pourront le faire que dans les conditions prévues par un décret pris en Conseil d'État.

des « anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » aux articles 4 et 7, puis du « président du conseil départemental d'Alsace » à l'article 5 et des « conseillers départementaux » de la CEA à l'article 8. La CEA est vraiment un département ! Or je ne pense pas que les Alsaciens aient voulu la disparition de leurs départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au profit d'un autre, fût-il dénommé Collectivité européenne d'Alsace. En outre, attendons-nous à des divisions internes, mes chers collègues parlementaires alsaciens, au sein de ce nouveau département, ne serait-ce que pour le choix de son chef-lieu. Je nous je rappelle que dans quatre sondages successifs réalisés en trente mois, plus de 80 % des Alsaciens ont indiqué vouloir sortir du Grand Est et retrouver une région Alsace avec toutes les compétences régionales. On est loin du compte

Quant à la possibilité pour la CEA de se voir déléguer par le conseil régional l'octroi de certaines aides économiques aux entreprises, ne rêvons pas ! Bien sûr, certains se consolent et pensent qu'il s'agit d'un premier pas, qui sera suivi par d'autres. Je ne suis pas de cet avis : si le Gouvernement avait voulu aller plus loin, il pouvait le faire à droit constant, notamment en constituant une collectivité à statut particulier. Par en cas de révision constitutionnelle instaurant un droit à la différenciation, pourquoi le Gouvernement irait-il plus loin, dès lors qu'il a répondu à ce qu'il appelle le « désir d'Alsace » en instaurant la CEA ? En conclusion, pour toutes ces raisons, ce texte ne me satisfait en aucun cas et, comme en première lecture, je voterai contre.

vote. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j'avais voté pour ce texte, tel que nous l'avions amendé au Sénat. Nous sommes favorables à davantage de décentralisation. Nous voulons tous satisfaire le « désir d'Alsace » des Alsaciens. Nous voulons une République moins jacobine, moins rigide, faisant confiance au terrain au lieu de tout vouloir régenter depuis Paris. Par nos amendements, nous avions ouvert aux autres départements les mêmes droits qu'aux Alsaciens, d'ailleurs avec le soutien des Alsaciens qui n'ont jamais demandé que l'on refuse aux autres ce qu'ils demandaient pour eux-mêmes. Or l'Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, a défait le travail du Sénat. Elle a même supprimé l'extension de l'écotaxe prévue en Alsace vers la Lorraine.

Autoriser l'écotaxe en Alsace et pas en Lorraine, c'est déporter tout le trafic de l'A35 vers l'A31. Injuste dans les principes, cette loi sera catastrophique dans les faits, du moins pour la Lorraine, c'est pourquoi, avec tous mes collègues lorrains,

Madame la ministre, considérant l'estime personnelle que je vous porte, j'aurais souhaité émettre avis favorable sur un texte qui devait répondre à un « désir d'Alsace

de consolidation du texte pour lui donner une charpente et une réalité. Le Gouvernement et, surtout, sa majorité à l'Assemblée nationale ont- hélas ! -préféré produire de la mousse, tout en faisant croire aux Alsaciens qu'ils leur servaient une vraie bière. Une forte communication positive n'effacera pas la réalité. En effet, dès l'article 1 A,

Je ne vais pas vous imposer la liste des insatisfactions : un chef de filât transfrontalier uniquement organisationnel, une charge routière non totalement une taxe de transit liée à une hypothétique ordonnance, un bilinguisme réduit à un enseignement complémentaire, toute une série d'ordonnances dont le contenu est ignoré au moment d'approuver ce texte Le mot Alsace reparaît, c'est un élément positif, mais cela constitue une faible avancée pour un texte sans relief, qui risque de générer autant de frustrations que de progression des autonomistes et des extrémistes. Vous en porterez la responsabilité, madame la ministre. Vous l'aurez compris, je m'abstiendrai sur ce texte.

l'on refuse à des départements qui sont exactement dans la même situation, ou à tout le moins dans une situation comparable, des demandes que l'on accorde à d'autres.

Vous l'aurez compris, mon vote sera négatif, mais je souhaiterais vraiment vous dire en quoi, à mon sens, le texte qui nous est présenté ne décline pas la déclaration de Matignon. Concernant le renforcement du bilinguisme, la déclaration de Matignon indiquait qu'« un nombre d'heures dédié à un apprentissage complémentaire, pratique et immersif de l'allemand pourrait être sanctuarisé dans l'emploi du temps des élèves de la maternelle au baccalauréat

la sanctuarisation dans l'emploi du temps des élèves ne me paraît pas compatible avec un enseignement facultatif ! C'est la raison pour laquelle j'affirme que, même si la lettre de la déclaration

temps des élèves. De même, la déclaration de Matignon précise que, pour soutenir la complémentarité des compétences entre l'État et les collectivités, « une nouvelle gouvernance devra être étudiée afin d'aller au-delà du dispositif de la convention quadripartite Le projet de loi indique désormais que la CEA crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande « qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées ». En quoi ce comité va-t-il au-delà

aurait été insupportable si l'autoroute A31, qui traverse la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, ne pouvait en bénéficier également. Il est regrettable que des députés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

Le Sénat a adopté. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique

d'offrir de nouvelles souplesses aux employeurs, tout en maintenant les garanties du statut général. Nous regrettons toutefois l'engagement de la procédure accélérée et des délais particulièrement contraints pour un texte qui dépasse aujourd'hui les 110 articles. Le projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 27 mars 2019 et voté en première lecture le 28 mai. Le texte issu des travaux du Sénat a été voté le 27 juin, et la CMP s'est réunie le 4 juillet. Nous l'aurons donc adopté définitivement en quatre mois. Nous espérons que les décrets d'application seront publiés avec autant de rapidité. Au Sénat, nous étions deux rapporteurs : Loïc Hervé s'est chargé des questions de déontologie, de formation, d'égalité professionnelle, et, pour ma part, je me suis concentrée sur les questions statutaires, le dialogue social et la discipline. Nous tenons à remercier nos collègues députés Émilie Chalas, rapporteure, et Guillaume Gouffier Cha, chef de file du groupe La République En Marche sur ce texte. Nous avons eu des échanges à la fois sincères et constructifs, qui se sont appuyés sur une connaissance pratique de la fonction publique territoriale et de la gestion des ressources humaines. Chacun a travaillé à un accord en engageant un dialogue direct et positif, même sur les points les plus techniques et en faisant les concessions nécessaires. Nous vous remercions également, monsieur le secrétaire d'État, de votre écoute et la qualité technique de vos interventions en séance publique, même si quelques divergences de vues subsistent entre nous. Je tiens à rappeler que le texte initial reprenait déjà plusieurs propositions du Sénat, comme l'harmonisation du temps de travail ou l'introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Lors de nos travaux, nous avons enrichi ce projet de loi en adoptant au total 154 amendements en commission et 125 amendements en séance publique. Le texte qui a été voté à une large majorité en commission mixte paritaire préserve de nombreuses avancées du Sénat. dont j'étais chargée, je mentionnerai six apports essentiels : le durcissement des règles applicables aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi pour éviter des situations sclérosées, qui coûtent cher aux collectivités la valorisation du mérite des agents, avec la possibilité d'attribuer des primes de service pour mettre en avant les résultats collectifs ; l'assouplissement du recours aux contrats dans la fonction publique territoriale, notamment pour les agents de catégorie C l'établissement d'une feuille de route triennale permettant aux employeurs territoriaux d'avoir plus de visibilité concernant les décisions en matière de ressources humaines de l'État, qui ont souvent un impact direct sur les budgets locaux l'amélioration des procédures disciplinaires, avec la suppression des commissions de recours ; enfin, la suppression du renvoi à un décret pris en Conseil d'État pour définir les missions des directeurs généraux des services. Sur ce dernier point, qui a fait couler beaucoup d'encre, nous invitons plutôt les différents acteurs à signer une charte de bonnes pratiques respectueuse du rôle des élus dans la gestion des ressources humaines. En parallèle, nous avons prévu de nouvelles garanties les DGS, comme leur exclusion du décret encadrant les recrutements dans les collectivités territoriales ou le renforcement des garanties offertes lorsqu'ils quittent leur poste. Nous ne sous-estimons pas les efforts consentis par l'Assemblée nationale, ce qui nous a conduits à accepter un texte de compromis. En contrepartie, plusieurs concessions importantes ont été nécessaires. Le point le plus délicat concernait les commissions administratives paritaires, les CAP. Notre rédaction commune acte la réduction du champ des CAP, même si nous ne sommes pas convaincus de l'opportunité de cette réforme. Pour améliorer le dispositif, nous avons toutefois prévu l'intervention d'un collège employeur dans les centres de gestion. En outre, nous avons admis la suppression de plusieurs articles concernant notamment le droit de réserve ou le licenciement pour insuffisance professionnelle après passage en CAP. Enfin, nous avons accepté que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnances pour réformer le dialogue social, alors qu'un projet de loi spécifique nous semblait préférable. Enfin, je tiens à remercier le président de la commission des lois, qui a, comme souvent, trouvé les mots justes pour faire accepter à Mme la rapporteure de l'Assemblée nationale la modification de l'article 28 apportée par notre collègue Michel Savin et des membres de tous les groupes de la commission des affaires culturelles du Sénat, afin d'éviter la remise en cause de la situation des conseillers techniques sportifs. Ainsi, mes chers collègues, les apports du Sénat étant substantiels, je vous invite à voter ce texte de compromis. Il permet de mieux répondre aux attentes des employeurs territoriaux, de mieux récompenser le mérite des agents et de mieux accompagner les personnes en situation de handicap, comme l'évoquera mon collègue Loïc Hervé,

avions affirmé avec constance notre volonté de parvenir à un accord avec l'Assemblée nationale sur ce projet de loi. C'est aujourd'hui chose faite, et nous nous félicitons de cet accord en commission mixte paritaire obtenu dans des délais tout aussi contraints que pour l'examen du texte lui-même. Il témoigne de la qualité des discussions entre nos deux assemblées et exprime la vitalité de notre bicamérisme. Je souhaite saluer les quelque 5,5 millions d'agents publics, qui oeuvrent chaque jour à l'organisation de nos services publics. À défaut de transformation en profondeur, il était à mon sens important d'apporter des améliorations qui sont aussi significatives qu'attendues par les agents et par les employeurs publics. Sur la réforme de la haute fonction publique, si l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances a finalement été rétablie, la volonté du Sénat de voir la création d'un tronc commun d'enseignements pour les agents publics de catégorie A a été respectée. toutefois rester vigilants sur ce point lors de la rédaction, puis de la ratification de ces ordonnances. En matière de déontologie, plusieurs avancées émanant du Sénat

a également été entériné. Je salue la sagesse de la commission paritaire qui a choisi de maintenir cette contribution majeure du Sénat. En contrepartie, nous avons accepté, notamment, la nomination par le Gouvernement de deux personnalités qualifiées au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la réduction du périmètre de contrôle systématique par cette dernière des

quant à son efficacité en l'état. Notre vigilance devra désormais s'exercer dans le cadre de notre fonction de contrôle. Je souhaiterais également évoquer les mesures d'accompagnement des agents publics en situation de handicap,

la modernisation du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, et de la consultation des associations représentant les personnes handicapées. En revanche, à mon grand regret, le principe d'un

paritaire a préservé des apports substantiels du Sénat, qui portent sur les droits et obligations des agents de la fonction publique. Le texte de compromis prévoit ainsi un meilleur encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale, pour éviter les grèves perlées et lever les freins à la continuité des missions de service public. Il prévoit la mise en oeuvre d'un entretien de carrière pour les métiers pénibles, ainsi que des dérogations à la formation obligatoire pour les policiers et les gendarmes, qui sont intégrés par voie de détachement dans la police municipale en raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. Ce texte consacre aussi de nouveaux droits pour les agents publics le congé de proche aidant, le télétravail ponctuel et le droit à l'allaitement. Telles sont les principales dispositions sur lesquelles je souhaitais faire le point. Elles sont le fruit d'une large concertation avec les représentants des élus et des agents publics. La parole

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de vous retrouver après que la commission mixte paritaire du 4 juillet dernier

Sur de nombreux points, l'apport de votre assemblée a été substantiel. De nombreuses dispositions ont été adoptées ici et contribueront à la réussite du projet que nous défendons en matière de fonction publique, Gérald Darmanin et moi-même pour la fonction publique d'État, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu pour la fonction publique territoriale et Agnès Buzyn pour la fonction publique hospitalière.

à l'élargissement du recours au contrat sur les emplois de catégorie C, ou encore à la prise en compte des objectifs collectifs du service dans la rémunération dite « au mérite » des agents territoriaux. Le Sénat est aussi à l'initiative de la création du congé de proche aidant pour les agents publics, de la création d'un entretien de carrière pour les agents exposés à des risques d'usure professionnelle, professionnelle, du renforcement de la place du recrutement sur titre dans la fonction publique territoriale. Je pense aussi à la mise en place d'un service minimum dans certains services publics territoriaux, en complément des règles déjà applicables dans les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, sans s'y substituer. Les SDIS bénéficient en effet de la possibilité, reconnue par la jurisprudence, d'encadrer le droit de grève des sapeurs-pompiers pour garantir la continuité du service et le respect de l'effectif minimum prescrit par le code général des collectivités territoriales en fonction des missions imparties.

l'encadrement du dispositif de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi dans la fonction publique territoriale- madame le rapporteur, je sais combien vous étiez attachée à ce que nous puissions avancer sur ce dossier -, ou encore le renforcement des droits des agents en situation de handicap, avec la portabilité des aménagements de poste et de leurs parcours professionnels, et l'expérimentation d'un dispositif dérogatoire d'accès à la fonction publique

Les autres dispositions seront applicables, pour l'essentiel, à compter du 1janvier 2020 ou dans le courant de l'année 2020. Pour respecter cet objectif, j'ai d'ores et déjà demandé à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique de travailler avec les deux directions générales compétentes pour les versants territorial et hospitalier

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la fonction publique est au coeur de notre vie démocratique, mais aussi des attentes de nos concitoyens. Ceux-ci les ont d'ailleurs vivement exprimées lors du grand débat une plus large intervention publique et un retour à des services publics de proximité, mais sans augmentation de la pression fiscale. Ces demandes font ainsi de l'avenir de la fonction publique un véritable défi. Ce projet de loi, qui n'est qu'une première étape, a pour objectif de transformer la fonction publique, sans en renier pour autant les fondements issus des lois statutaires de 1946 et de 1983. Il vise à mettre en oeuvre les moyens indispensables à sa modernisation, en portant une série de modifications, souvent techniques, dans trois domaines essentiels : tout d'abord, la simplification du dialogue social et les nouveaux outils managériaux l'élargissement du recours aux contractuels ; enfin, le renforcement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je me félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un texte de compromis grâce aux apports du Sénat. apports du Sénat. Je me réjouis tout particulièrement que le travail au Sénat ait permis de mieux répondre aux attentes des employeurs locaux. En effet, notre assemblée a donné de nouveaux outils aux employeurs territoriaux, notamment pour lutter contre les grèves perlées qui perturbent le bon fonctionnement des services publics. Le Sénat a également donné plus de prévisibilité aux élus locaux en obligeant l'État à publier une feuille de route triennale, dans laquelle il préciserait les incidences financières de ses décisions en matière de ressources humaines sur les budgets locaux. Je suis heureux que le texte permette de renforcer les obligations des fonctionnaires territoriaux momentanément en recherche d'emploi, tout en améliorant leur accompagnement pour un retour vers l'emploi. de loi mettra ainsi fin à des situations qui n'étaient bénéfiques ni pour les agents ni pour les employeurs. Je me réjouis aussi que notre assemblée ait amélioré les procédures disciplinaires en supprimant les commissions de discipline de recours, l'agent pouvant toujours contester sa sanction devant un juge administratif. Enfin, je suis satisfait que le Sénat ait assoupli le recours aux agents contractuels, notamment pour ceux de tout en renforçant leur formation. De même, il a facilité le recrutement des agents titulaires d'un diplôme d'État et allégé les obligations de formation des policiers municipaux lorsqu'ils sont anciens gendarmes ou policiers. ou policiers. Je me félicite que le texte élaboré par la commission mixte paritaire comporte plusieurs avancées importantes du Sénat qui visent à mieux récompenser le mérite des agents et à leur garantir de nouveaux droits. Parmi ceux-ci, je tiens à souligner la création d'un entretien de carrière pour les métiers les plus pénibles, l'extension du congé de proche aidant, le télétravail ponctuel et le droit à l'allaitement. Je souhaite également mettre l'accent sur les apports de notre assemblée qui permettront de mieux accompagner les personnes en situation de handicap. En effet, je me réjouis que le texte permette, non seulement de généraliser les référents handicap et d'autoriser la titularisation des apprentis handicapés,

rare, équilibrée, qui mérite d'être confortée et soutenue à l'avenir. Les deux assemblées ont travaillé de concert pour consolider et compléter les dispositions initiales de ce texte, notamment grâce à l'adoption de plusieurs centaines d'amendements lors de son examen en commission et en séance publique.

qui a présidé lors de nos échanges procède, il faut le rappeler, de la méthode insufflée par le secrétaire d'État, Olivier Dussopt. Ce texte est aussi le fruit d'une grande concertation, menée très en amont, avec les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des collectivités locales et des employeurs hospitaliers. Réformer les règles applicables aux 5,5 millions d'agents du service public sans préjudice des lois statutaires n'était pas une mince affaire : le défi est relevé. Le projet de loi répondait à cet enjeu indispensable de modernisation de la fonction publique, au travers de cinq titres. adapter et renforcer le dialogue social dans la fonction publique à travers notamment la mise en place des futurs comités sociaux. La création du rapport social unique représente également un nouvel outil de pilotage des ressources humaines. Si la réforme des commissions administratives paritaires a parfois suscité le débat, nous sommes arrivés à une position de compromis, grâce notamment aux propositions du Sénat. Le titre II qui porte sur les leviers managériaux a été considérablement consolidé par nos deux assemblées. Je me réjouis à mon tour du renforcement des obligations de formation au bénéfice de l'ensemble des agents publics. Enfin, je me félicite du consensus trouvé autour de l'article 10 , afin d'introduire une prime de précarité pour les contrats d'une durée inférieure à un an, notamment dans la fonction publique hospitalière. Nous mettons fin à une inégalité entre secteur public et secteur privé, qui n'était pas justifiée. En ce qui concerne les questions de transparence, nous pouvons être

Concernant l'habilitation prévue à l'article 22, nous avons abouti à une rédaction plus précise, tout en laissant une latitude suffisante pour permettre à la mission de M. Frédéric Thiriez

Le Sénat a enrichi ce projet de loi en adoptant, au total, 154 amendements en commission et 125 amendements en séance publique. Nous avons travaillé en fonction de la pertinence des propositions

nous ne sommes pas surpris, tant les convergences sont grandes entre la majorité sénatoriale et la majorité présidentielle pour briser le modèle social de notre pays, en affaiblissant la puissance publique au profit des intérêts privés ... C'est exactement l'objet du projet de loi.

et qui, par leur esprit de responsabilité, pallient tous les dysfonctionnements pour garantir la continuité du service public. Nous pensons bien au contraire qu'au lieu d'accabler et de vouloir faire passer ces fonctionnaires pour des sortes de privilégiés, vous feriez mieux de vous intéresser à ce qu'ils vous disent. vous aussi, monsieur Bas ! N'entendez-vous pas, par exemple, ces urgentistes en grève depuis plusieurs semaines qui vous disent qu'ils n'en peuvent plus, que c'est dangereux et qu'il va y avoir non-assistance à personne en danger ? Vous ont-ils demandé l'instauration de saisonniers dans la fonction publique hospitalière ? Pas du tout, ils demandent de la stabilité et des moyens supplémentaires ! N'entendez-vous pas ces personnels de l'éducation nationale qui vous alertent sur l'école inégalitaire que vous êtes en train de bâtir ? Ne voyez-vous pas le mal-être de ces agents qui ne trouvent plus de sens à leur mission, alors qu'on leur demande de faire toujours plus avec moins, de ces fonctionnaires qui voient les conséquences dramatiques de la dégradation du service public décidée au plus haut niveau et devant laquelle ils sont impuissants ? Ne voyez-vous pas, enfin, les difficultés de ces fonctionnaires qui touchent dont les conditions de vie sont toujours plus difficiles, notamment en raison du gel du point d'indice ? Non, manifestement, vous ne les entendez et ne les voyez pas, car vous êtes trop occupés à satisfaire les intérêts de ceux qui savent se faire entendre de votre majorité : les lobbies, les grandes entreprises, les exilés fiscaux, les vrais privilégiés en somme, ceux qui ont intérêt à rendre confus le sens de l'action de la puissance publique. Dans ce cadre, les quelques avancées du texte en matière de déontologie sont de simples trompe-l'oeil, puisque la porosité entre le public et le privé sera renforcée, tout comme les pratiques de pantouflage et de rétropantouflage. On verra bien si l'histoire nous donne tort. Ce projet de loi s'inscrit incontestablement dans une démarche cohérente. Vous bradez les biens publics qui sont le patrimoine de tous. Vous libéralisez les services publics pour permettre à vos amis de faire des profits, et, maintenant, vous remplacez les fonctionnaires par des contractuels, afin « de promouvoir la diversification des viviers de recrutement », comme si ces hommes et ces femmes étaient de vulgaires poissons d'élevage ! Vous poursuivez votre casse des outils de l'égalité républicaine. Eh oui, les fonctionnaires sont bel et bien les outils privilégiés de l'égalité républicaine, garantie par la loi. Pour ce faire, notre modèle républicain a permis l'émergence d'une fonction publique de carrière, donc du temps long, fondée sur les notions d'égalité, de responsabilité et d'impartialité. Ce modèle visait à garantir l'accès aux services publics à l'ensemble de nos concitoyens et en tout lieu.

soumis aux aléas des jeux politiques, puisqu'ils seront très directement employés par l'autorité politique. Nous craignons non seulement le retour de l'arbitraire et du clientélisme, mais également le retour du fonctionnaire sujet, rouage de l'administration, contre lequel le statut s'est construit. Votre projet, au fond, revient à faire disparaître l'État

mal. Tout de même ! Pour le reste, toutes les aggravations ont été maintenues, notamment les attaques contre le droit de grève. Après la remise en cause du rôle des commissions administratives paritaires, voilà un nouvel exemple du peu de cas que vous faites du dialogue social et des droits fondamentaux. ce projet de loi favorise une précarité accrue par un recours étendu aux futurs contrats de projet, qui concerneront demain l'ensemble des catégories de la fonction publique. Il s'agira de fonctionnaires de seconde zone pour un service de seconde zone, qui justifiera demain la privatisation de pans entiers de service public. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce texte qui organise le dépérissement de la fonction publique et la captation de l'appareil d'État par les intérêts privés, en détournant de l'intérêt général les finalités de l'action publique. Tout ce qui est excessif

portent un regard nuancé sur la version finale d'un projet de loi issu d'un compromis entre la majorité de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Il serait pourtant incorrect de ne pas rappeler que le projet de loi avait été profondément amélioré après son passage au Sénat en première lecture. C'est la preuve que la droite sénatoriale avait su faire preuve d'écoute à cette occasion. Nous sommes déçus de ne pas avoir trouvé la même oreille du côté de La République En Marche, ce qui explique que plusieurs des avancées défendues en séance par les sénateurs socialistes soient absentes du texte de la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire a toutefois conservé deux de nos apports importants, à savoir l'exclusion des conseillers techniques sportifs du détachement d'office et le contrôle de la HATVP lorsque les collaborateurs de l'Élysée et les membres de cabinets ministériels créent une entreprise en cas de pantouflage et de rétropantouflage.

la définition des centres des intérêts matériels et moraux par décret ; le recouvrement automatique des sommes dues par un fonctionnaire qui n'a pas honoré son engagement de servir ; l'interdiction par les représentants d'intérêts d'exercer toute action pour le compte ou auprès d'une personne morale de droit public, dont ils ont été l'agent public au cours des trois dernières années l'allongement à dix-huit mois du délai laissé aux employeurs pour négocier la durée du temps de travail ; l'évaluation à mi-parcours de l'expérimentation de la rupture conventionnelle ; enfin, la suppression du caractère obligatoire de la pénalité financière pour défaut d'élaboration d'un plan d'action d'égalité professionnelle entre femmes et hommes-

et du recours au contrat sur les emplois permanents de la fonction publique territoriale ; une version de la prime de précarité réduite à la portion congrue, puisque les plus précaires des contrats de la fonction publique hospitalière en sont exclus ; la restriction du droit de grève dans la fonction publique territoriale ; la cessation de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi au bout de cinq ans

Nous voterons donc contre ce projet de loi, d'ailleurs rejeté par les organisations syndicales représentatives de la fonction publique. M. Vallaud a rappelé à l'Assemblée nationale que nous sortions de la longue histoire de la fonction publique avec ce texte. Permettez-moi d'ajouter que vous imposez ce tournant dans un contexte social pourtant difficile. Alors que M. le secrétaire d'État a confirmé le gel du point d'indice, nos inquiétudes persistent sur la manière dont le dialogue social pourra pourra être mené avec les reculades que comporte ce texte. La santé au travail et les risques professionnels seront relégués au second plan avec la suppression des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La transparence des évolutions de carrière ne sera plus assurée,

entre salariés du privé couverts par une mutuelle et fonctionnaires. Ce jour de carence pour le public n'était-il pas supposé instaurer l'égalité entre les salariés du public et du privé ? Ce nivellement par le bas sur les absences de courte durée illustre bien la tendance à l'oeuvre aujourd'hui. En outre, je crains que nous ne vivions la même histoire avec la réforme des retraites les fonctionnaires titulaires et contractuels ne semblent pas sauter au plafond à l'annonce de cette réforme à venir, ou alors il s'agit de manifestations de soutien qui m'ont échappé. Cette réforme bénéficiera-t-elle aux employeurs publics ? Si certaines mesures faciliteront leur quotidien, je crains que, très vite, nous ne regrettions le peu de progrès sociaux que cela entraînera pour la fonction publique en termes d'attractivité. Votre philosophie est de privilégier le recours aux contractuels pour répondre à des besoins qui sont, selon vous, trop difficiles à satisfaire à cause de l'inertie supposée de la fonction publique. Mais ce faisant, vous courez le risque de faire perdre à la fonction publique l'un de ses principaux avantages concurrentiels ses agents. J'aime à rappeler cet exemple, relevé par la presse, d'une SNCF qui peine à attirer des candidats aux postes les plus exposés à la concurrence en termes de recrutement. Il ne suffit pas de rappeler les vertus supposées d'une nouvelle culture managériale pour compenser cette faiblesse. chers collègues, nous rejetons cette réforme de la fonction publique dont les effets délétères se feront probablement sentir sur le long terme. Ce gouvernement supprime sans doute moins de postes de fonctionnaires que ne l'aurait souhaité M. Fillon,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'heure du bilan du travail parlementaire accompli lors de ces quelques mois d'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique, je tiens, tout d'abord, à souligner l'extrême efficacité de notre procédure législative. Entre son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale le 27 mars dernier et notre vote d'aujourd'hui, quatre mois ont suffi pour parvenir à un compromis transpartisan sur des sujets aussi sensibles que l'encadrement du droit de grève, la réforme des commissions administratives paritaires ou l'encadrement du temps de travail. Si certains d'entre nous y voient de la précipitation, notre groupe en fait une tout autre lecture, en considérant que ce texte donne force de loi à des propositions restées en souffrance pendant plusieurs années. Il suffit de relire les comptes rendus des auditions de commission ou le compte rendu de la séance pour en prendre conscience. À l'Assemblée nationale comme ici, à l'image de notre représentativité, les points d'opposition sont connus depuis longtemps le poids des syndicats dans la fonction publique, l'articulation entre un statut de la fonction publique territoriale et l'autonomie des collectivités, l'équilibre entre les droits et les obligations des agents, ou encore le périmètre de leur statut. En réalité, la question reste toujours la même : quelle forme donner à l'État pour qu'il satisfasse les besoins de nos concitoyens ? « Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un État plus ramassé, mais plus efficace dans l'accomplissement des missions qui sont les siennes »

Il faut donc saluer notre rigueur collective, qui nous a conduits à ne pas laisser errer davantage nos débats sur des sujets pour lesquels nous connaissons ô combien la position des uns et des autres et à nous concentrer sur des problématiques qui nécessitaient un consensus. C'est le cas du contrôle de déontologie pour les mobilités entre les agents du secteur privé et du secteur public. Dès lors que l'on encourage davantage ces mobilités, notamment depuis la loi du 3 août 2009, il fallait nécessairement adapter un dispositif qui avait été pensé au moment où celles-ci avaient vocation à rester marginales. Il est clair que, depuis 1983 et, plus encore, depuis 1946, les parcours professionnels des Français ont évolué en s'allongeant et en se diversifiant. La fonction publique ne peut rester hermétique à ces changements, et c'est pourquoi, au sein du groupe du RDSE, nous avons toujours défendu une approche pragmatique en la matière : autoriser les mobilités tout en prévenant les conflits d'intérêts. Le système finalement retenu devrait permettre de simplifier la vie de la majorité des agents souhaitant se reconvertir professionnellement, à l'exception de « ceux dont la nature ou le niveau de fonction le justifient

-, notamment l'inscription d'un contrôle en cas de réintégration d'un fonctionnaire et la publicité de la HATVP. Nous verrons à l'usage si les sanctions prévues et la composition du nouveau collège permettent de mettre fin aux travers attribués à la commission de déontologie. Alors que, en 1983, on débattait de la suppression de la catégorie D, ce sujet déontologique a fait émerger la question de la reconnaissance d'une catégorie A+. Nous pensons qu'une telle reconnaissance serait opportune, dès lors qu'elle concernerait les catégories d'emploi les plus proches du pouvoir politique, afin d'appliquer à celles-ci des règles spécifiques. Enfin, le maintien d'une obligation de documenter le phénomène de pantouflage et l'obligation de remboursement de frais de scolarité à l'article 16 constituent une première étape dans la restauration de la force de l'engagement décennal. Je voudrais également souligner quelques avancées en matière sociale : une meilleure prise en compte du handicap des agents publics, pour laquelle le Sénat a fourni un travail décisif, mais également certaines évolutions législatives destinées à améliorer l'articulation entre vie de famille et vie professionnelle pour les femmes et adapter les avantages familiaux à la nouvelle fragilité des couples. Sur ce dernier point, je fais référence à l'adaptation du supplément familial de traitement, introduite sur notre initiative, qui devrait contribuer à apaiser les relations financières après la séparation d'un couple d'agents publics. Nous retenons par ailleurs des avancées contrastées selon la fonction publique concernée. Dans la fonction publique territoriale, les avancées sont considérables pour les employeurs locaux, grâce au maintien par la CMP des apports du Sénat dans un texte déjà imprégné de la sensibilité du secrétaire d'État à ces sujets. Nous espérons que le texte permettra de faciliter le recrutement d'anciens agents du ministère de l'intérieur dans les rangs des policiers municipaux, un sujet que j'avais soulevé dès l'examen en commission. Concernant la fonction publique hospitalière, nous retenons également quelques avancées, telle que la création d'une prime collective, bien que la situation de départ soit particulièrement dégradée. Concernant la fonction publique d'État, enfin, les portées des modifications introduites sont les plus difficiles à anticiper et divisent les membres de notre groupe. Pour certains d'entre nous, la marginalisation des commissions administratives paritaires, ou CAP, et les mesures visant à renforcer le recours aux contractuels menacent à terme le statut. D'autres y voient au contraire des moyens de revitaliser une machine étatique, par la diversification des modes de recrutement et le renforcement de la notion de carrière, qui peuvent s'avérer être un moyen de sauver le statut. Ces derniers considèrent pour autant qu'une attention particulière doit être portée aux risques de précarisation des contractuels, qui sont finalement les plus vulnérables de nos agents publics. Dans l'attente que l'avenir infirme ou confirme ces dernières observations,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, mon intervention se limitera à l'alinéa 11 modifié de l'article 28. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la commission des lois

alinéa que le Sénat avait adopté un amendement porté par l'ensemble des groupes politiques. Ce dispositif retenu par la Haute Assemblée vise à exclure les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport d'un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives. Le texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale a fait l'objet d'une controverse n'ayant échappé à personne. En effet, le mouvement sportif y a vu un moyen détourné de forcer le détachement automatique des conseillers techniques sportifs, ou CTS, auprès des fédérations. Ses acteurs se sont donc sentis trompés par le Gouvernement, car l'adoption de l'alinéa en question est intervenue alors même que des discussions venaient d'être entamées au sujet de l'avenir des CTS entre les fédérations, les syndicats et le ministère des sports. Je tiens à rappeler ici que les CTS occupent une place unique dans l'organisation du sport français. Ils ont contribué à faire de la France l'un des pays ayant le plus développé des politiques de sport de haut niveau et de sport pour tous. Ils sont au coeur du modèle sportif français, qui s'est construit à partir des années 1960 autour des structures associatives- les fédérations sportives agréées -, d'une part, et du ministère des sports, d'autre part, chargé d'apporter une expertise sous la forme d'une mise à disposition de personnels qualifiés. Le rôle joué par les CTS est d'une importance d'autant plus capitale que la France s'apprête à participer aux jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020 et à organiser ceux de Paris en 2024. Ces échéances appellent une mobilisation de tous. Par ailleurs, nous avons entendu les craintes des petites fédérations, qui se trouveraient particulièrement menacées par le détachement automatique. Faute de moyens financiers et de ressources humaines, elles auraient effectivement beaucoup de difficultés à faire face à une situation de désorganisation totale. Aussi, la prégnance des CTS au sein du système sportif français rend inconcevable ce transfert automatique, voulu de force par le Gouvernement. L'adoption de notre dispositif a pour objectif, monsieur le secrétaire d'État, de rétablir un climat propice à une discussion apaisée et de redonner confiance aux acteurs du monde sportif, afin que des négociations sereines sur l'avenir des CTS soient ouvertes. Dans cette réflexion, il ne faudra pas non plus oublier le cas des conseillers d'animation sportive et des formateurs qui, eux aussi, jouent un rôle important. Nous avons pu constater que la ministre des sports avait nommé, pour répondre à cette crise, deux tiers de confiance qui doivent rencontrer l'ensemble des acteurs concernés et remettre un rapport contenant des préconisations à l'automne. Nous sommes bien conscients que le n'est pas souhaitable concernant le CTS : se pose la question de leur nombre, de leur formation, de leur répartition au sein des fédérations et de leurs missions entre la haute performance et le développement des politiques publiques, comme le sport santé, le handisport, le sport à l'école, le soutien au sport féminin, le renforcement des actions d'information et de prévention sur la violence, le racisme, l'homophobie, etc. Toutes ces missions, qui constituent de véritables enjeux de société, doivent être au coeur des discussions. Nous en sommes tous convaincus, le sport tient un rôle important en termes de santé publique, de solidarité, d'intégration et de partage ; il a aussi une place considérable dans l'économie de notre pays. En fait, les questions qui se posent aujourd'hui sont bien de savoir quelle place on lui donne au sein des politiques publiques. Le Gouvernement prévoit une grande loi sur le sport pour le premier trimestre de 2020. Il reste donc quelques mois à la ministre pour trouver un accord et intégrer, dans cette future loi, la nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement des CTS. C'est donc avec une certaine confiance dans la réussite de ces évolutions, nécessaires pour le développement de la pratique sportive dans notre pays, que nous voterons ce texte. La parole est à M. Michel Canevet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord, au nom du groupe Union Centriste,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, madame, monsieur les rapporteurs de la commission des lois, mes chers collègues, ce projet de réforme de la fonction publique est le fruit du travail conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat. Examiné selon la procédure accélérée, le texte a été enrichi

première lecture au Sénat, près de 1 030 amendements ont été déposés et 279 adoptés. C'est sur cette base que la CMP a été conclusive. Ainsi, cette loi instaure des « lignes directrices de gestion », relevant plus d'une « évolution » que d'une transformation. Les apports du Sénat, substantiels, permettront de mieux répondre aux attentes des employeurs territoriaux, de mieux récompenser le mérite des agents et de mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Apparaissent dans la fonction publique des outils du privé : la rupture conventionnelle sera expérimentale pendant cinq ans pour les fonctionnaires. De même, des dispositifs que des associations d'élus locaux réclamaient sont introduits : la rémunération au mérite collectif, la procédure disciplinaire révisée et la limitation du droit de grève dans les collectivités.

A également été adopté au Sénat et confirmé en CMP un outil qui déterminera la stratégie pluriannuelle de la collectivité en matière de ressources humaines : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec des orientations générales pour la promotion et la valorisation des parcours. La question de l'apprentissage dans la fonction publique a également été au coeur des débats. L'apprentissage est un outil essentiel de l'insertion des jeunes, auquel je suis particulièrement attentive, notamment dans j'en suis heureuse -l'amendement du Gouvernement visant à aligner le coût de l'apprentissage dans la fonction publique par rapport au secteur privé. Cela ne fait pas obstacle au versement d'une majoration de rémunération, dans des conditions qui seront précisées par décret. Le Sénat, garant de la situation financière des collectivités territoriales, a favorisé le financement de l'apprentissage dans les collectivités, grâce à l'intervention de notre collègue Françoise Gatel. Ce financement sera pris en charge par le CNFPT à hauteur de 30 par l'État à hauteur de 40 %, soit un montant de 31 millions d'euros. Le reste à charge sera assumé par les employeurs territoriaux, sachant que les collectivités, dont la situation financière est très tendue, n'embaucheront pas de jeunes en apprentissage si le coût demeure trop élevé.

L'excellent travail, porté avec conviction par les rapporteurs de la commission des lois, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, nous permet d'aboutir, dans un temps record, à un texte équilibré, répondant à une réalité et un besoin.

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

visant à assurer notre souveraineté nationale et lutter contre le pantouflage et le rétropantouflage. La porosité, très prégnante, est effectivement de plus en plus avérée entre la haute fonction publique et certaines entreprises extra-européennes, qui

l'examen des comptes de l'année 2018, et malgré l'adoption de chacun des articles, le Sénat a choisi de ne pas adopter le projet de loi de règlement qui lui était soumis. Nous nous en sommes étonnés au sein du Gouvernement, considérant que la loi de règlement n'est qu'un exercice de constatation, un moment de vérité plus que de contradiction. Bien sûr, il pourrait y avoir matière à polémique si la sincérité des comptes présentés au Parlement était sujette à caution, mais vous aviez vous-même souligné, monsieur le rapporteur général, l'effort de sincérité inédit caractérisant ce texte, comme l'avait fait avant vous le Haut Conseil des finances publiques. L'exercice

Constatons aussi que, l'année dernière, le ratio de dépenses publiques est passé de 55 % à 54,4 % du PIB, crédibilisant notre objectif de baisse de 3 points sur le quinquennat. Constatons encore que, l'année dernière, le taux de prélèvements obligatoires a diminué de 0,2 point de PIB, pour s'établir à 45 % du PIB. Constatons enfin que, l'année dernière, le résultat patrimonial de l'État a été négatif de 51,9 milliards d'euros, soit le meilleur résultat depuis 2008, et la dette publique s'est stabilisée à 98,4 % du PIB, ce qui n'était pas arrivé depuis des années.

; il n'a pas seulement tiré parti de la croissance. Les efforts en dépenses sont bien réels, avec un déficit inférieur de près de 10 milliards d'euros à la prévision en loi de finances initiale et une sous-exécution de 1,4 milliard d'euros par rapport à la norme de dépense.

vous serez certainement rassurés. En effet, le Gouvernement, sans renoncer à son objectif de baisse de la dépense publique de 3 points de PIB, financera en même temps la plus forte réduction d'impôts depuis quarante ans- plus de 27 milliards d'euros, avec la suppression de la taxe d'habitation ou encore la baisse de l'impôt sur le revenu

J'ai, devant l'Assemblée nationale, salué les avancées réalisées dans le cadre du « printemps de l'évaluation », ainsi que les efforts entrepris pour doter les députés de moyens de contrôle et d'évaluation indépendants. Mais je n'ignore rien des évolutions qui sont en cours ici, singulièrement au sein de votre commission des finances. Vos travaux de contrôle ont montré leur utilité. Je pense par exemple à vos propositions en matière de TVA sur le e-commerce, élaborées de manière transpartisane, et qui ont éclairé le Gouvernement dans la préparation du « paquet » de mesures en matière de TVA que nous proposerons en projet de loi Je pense aussi à la mobilisation de la commission des finances pour disposer du « code source » de l'impôt : le simulateur d'impôt sur le revenu mis en ligne la semaine dernière sur le site du ministère de l'action et des comptes publics devrait vous donner satisfaction, tout comme la publication en open data de plusieurs jeux de données fiscales. Il faut certainement aller plus loin, et je sais que le Parlement, ici comme à l'Assemblée nationale, saura relever le défi. Ces encouragements de la part du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, sont à la fois sincères et intéressés : sincères, parce que nous sommes tous ici d'accord sur l'objectif, à savoir faire des débats budgétaires un exercice plus transparent, plus informé, donc plus démocratique ; intéressés, parce que nous espérons que ces nouveaux outils d'évaluation et de contrôle vous permettront à l'avenir de reconnaître la bonne exécution de nos priorités politiques et, qui sait, peut-être, de mieux les partager. La parole est

le projet de loi de règlement constitue aussi le résultat concret de la politique fiscale et budgétaire menée par le Gouvernement. C'est à ce titre- nous ne sommes pas simplement des comptables, comme le serait la Cour des comptes -qu'il est soumis à l'approbation du Parlement. Et c'est dans ce cadre que le Sénat a décidé de ne pas l'adopter. Pour quelles raisons ? L'explication essentielle tient au fait que le Gouvernement a pu disposer, une nouvelle fois, d'une croissance supérieure à son potentiel et d'un fort dynamisme des prélèvements obligatoires,

! Ensuite, contrairement à ce que le Gouvernement indique, il n'y a pas eu de baisse de la dépense publique en volume. Si l'on neutralise les facteurs exceptionnels- Areva, taxe à 3 % -et que l'on prend en compte les crédits d'impôt enregistrés en dépense,

tandis que les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale confortent leurs excédents, l'État, au contraire, voit son déficit se creuser de plus de 8 milliards d'euros par rapport à 2017, pour atteindre 76 milliards d'euros en 2018.

l'année 2018 a également constitué une année d'application d'une politique fiscale et budgétaire dont le Sénat n'a pas soutenu plusieurs de ses mesures emblématiques, pour des raisons que je ne rappellerai pas ici. Voilà brièvement présentées les principales critiques formulées quant à l'exécution du budget de l'année 2018.

et de ne pas reporter les efforts qui pourraient être réalisés de façon raisonnable, sans porter atteinte à la croissance ni renoncer aux marges de manoeuvre qu'offre indéniablement la période actuelle de taux bas pour soutenir l'investissement.

Nous avons voté l'article liminaire, qui présente le solde structurel et solde effectif de l'ensemble des administrations publiques. Nous avons entériné la tenue des finances publiques par rapport à l'autorisation en loi de finances initiale le déficit public est ainsi amélioré de 0,3 point de PIB par rapport à la prévision de la loi de finances initiale. Nous avons voté l'article 1, qui présente les résultats du budget de l'année 2018, savoir l'amélioration du solde budgétaire de l'État et la maîtrise des dépenses en dépit d'une révision à la hausse de la charge de la dette et du prélèvement sur recettes, au profit de l'Union européenne. Nous avons voté l'article 2, qui présente le besoin de financement et les ressources de financement pour l'année ; l'article 3, qui retrace le compte de résultat de l'exercice 2018 ; l'article 4, qui régularise les dépassements constatés et procède à l'annulation des crédits non consommés ni reportés ; l'article 5 sur les budgets annexes ; l'article 6 sur les comptes spéciaux. Nous avons voté l'article 7, qui procède à la ratification de deux décrets, ainsi que l'article 8. Le Sénat a donc voté chacun des articles du texte .... Mais il a finalement rejeté l'ensemble de celui-ci ! C'est une décision politique ! La semaine passée, tous les orateurs ont introduit leur propos relatif au projet de loi de règlement et au débat d'orientation des finances publiques en rappelant qu'il s'agissait de regarder à la fois vers le passé, en débattant l'exécution de l'année 2018, et vers l'avenir, en débattant de la stratégie des finances publiques de notre pays. je dois vous le dire, mes chers collègues, au regard de la première lecture, nos concitoyens auront surtout eu, je crois, le sentiment de regarder vers le passé, un passé politique qu'ils souhaitent révolu. Ces choix politiques conduisant au rejet du texte au prétexte que le budget initial n'aurait pas été approuvé n'appellent que peu de discussion. Je me tournerai donc vers les mesures qui ont été annoncées et qui concernent les comptes de la Nation. Nous avons, grâce aux premiers documents budgétaires disponibles, les priorités du Gouvernement. Je citerai : le renforcement des mesures de lutte contre la pauvreté, notamment avec la montée en puissance du plan pauvreté ; la poursuite des investissements dans dans les fonctions régaliennes de l'État- je rappelle ici l'augmentation de 1,7 milliard d'euros par an pour les armées ; l'investissement dans le capital humain et la formation, avec l'augmentation de plus de 1 milliard d'euros pour 2020 des crédits de l'éducation nationale ; l'écologie, non seulement par la hausse des crédits, mais aussi par l'adoption d'un budget vert, c'est-à-dire que, pour la première fois, les décisions budgétaires seront analysées par rapport à nos engagements environnementaux et à l'accord de Paris. En parallèle, seront menés des chantiers de réforme majeurs pour notre pays, à la fois en termes d'équilibre de nos finances publiques et en termes de justice sociale. la réforme de l'assurance chômage pourra dégager des ressources nécessaires aux comptes de la Nation, tout en mettant en oeuvre le principe de justice. Elle permettra, par exemple, de stopper l'abus des contrats courts. Celle des retraites pourra clarifier l'organisation complexe des régimes et donner plus de liberté aux Français. Elle aura aussi pour conséquence des transferts entre les régimes qu'il faudra assumer par exemple des hommes vers les femmes, aujourd'hui lésées, ainsi qu'en faveur des familles monoparentales. Enfin, nous suivrons le chantier de la réorganisation de l'État dans les territoires, pour faire suite aux circulaires du Premier ministre du 24 juillet 2018 et du 5 juin 2019. Il doit permettre la simplification du paysage administratif avec une nouvelle déconcentration. Face à ces chantiers, nous devrons, mes chers collègues, nous rassembler et débattre pour un seul objectif : la réussite de notre pays. Le Gouvernement a envoyé des signaux forts, notamment aux élus que nous sommes.

conclure, notre groupe votera ce projet de loi de règlement. Nous espérons que la discussion du projet de loi de finances pour 2020 sera l'occasion pour les membres de notre assemblée qui voudront se tourner vers les Français de le faire collectivement.

L'analyse du budget 2018 montre que vous vous êtes évertué à continuer les baisses d'impôts sur les plus riches et sur les sociétés. Vous avez poursuivi la suppression de l'ISF- hop ! un cadeau de 3,2 milliards d'euros aux riches contribuables ; vous avez diminué le taux de l'impôt sur les sociétés, pour près de 1,2 milliard d'euros. Puis, vous lancez la première étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des foyers, qui a coûté 3 milliards d'euros. Enfin, vous instaurez prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, soit 1,6 milliard d'euros abandonnés à ceux qui touchent des revenus financiers. Tout cela, une fois de plus, au nom de la lutte contre le chômage ! Pourtant, un simple regard historique montre qu'offrir des cadeaux fiscaux aux plus riches ne fait pas reculer le chômage. Le taux marginal d'imposition sur le revenu et le taux d'imposition sur les sociétés sont en baisse quasi continue depuis 1986. À cette date, il était encore à 65 % pour l'impôt sur le revenu, tandis que le taux d'imposition sur les sociétés était de 45 %. 1986 a été le point de départ d'une baisse continue de l'imposition des contribuables les plus riches, la courbe du chômage, elle, n'a pas suivi le même chemin. Elle n'est jamais passée durablement sous le seuil des 9 d'alors. En fin de compte, les mêmes recettes conduisent aux mêmes résultats. Notre vote contre trouve ici sa première justification : le refus d'une politique qui, en définitive, subventionne de manière déguisée le chômage.

En 2018, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a vu son taux passer de 6 % à 7 %, ce qui a coûté à nos finances publiques 3,5 milliards d'euros. Et vous avez acté sa transformation en allégements de cotisations sociales : 3,5 milliards d'euros, qui s'ajoutent à presque 100 milliards d'euros. Cela restera dans l'histoire sociale, économique et financière Depuis 2013, on aura mis 100 milliards d'euros dans le CICE. Avec quel effet tangible sur l'emploi ? Soyons précis et concrets. Je voudrais confronter l'efficacité de ces mesures à la situation de l'emploi dans mon département du Val-de-Marne. Cette comparaison démontre le caractère passéiste et assez idéologique de votre politique. Les premiers allégements de cotisations sociales ont été lancés par M. Balladur- rendez-vous compte ! -, en 1993. Pourtant, entre 1989 et 2000, le chômage dans mon département est passé de 6,2 % à 7,2 %. Aucun effet positif, donc. Loin de s'arrêter, les cadeaux fiscaux ont continué : la ristourne dite « Juppé », lancée en 1996 et accentuée en 2003 sur l'initiative de M. François Fillon, a eu les mêmes effets Si bien que, à la moitié de la décennie, en 2005, dans mon département, le taux de chômage avait encore grimpé pour atteindre 8,3 %. Vous noterez que ces données excluent la crise économique. Une fois encore, mes chers collègues, il n'y a aucune efficacité des cadeaux fiscaux dans la lutte contre le chômage ! Voici la seconde raison pour laquelle nous nous opposons à votre politique fiscale. Aussi, je vous en conjure, il faut sortir des dogmes qui règnent depuis des décennies.

Ne croyez-vous pas qu'il puisse y avoir au moins une colère sourde et un sentiment d'injustice ? L'emploi est la première préoccupation des Françaises et des Français, et le chômage pénalise en premier lieu les jeunes et les femmes. Pourtant, en plus d'offrir des cadeaux fiscaux injustes et inefficaces, vous réduisez les moyens permettant de lutter contre le chômage, monsieur le secrétaire d'État. C'est la troisième raison pour laquelle nous nous opposons à votre politique.

Citons notamment la fin du recours à des décrets d'avance et l'amélioration de la prévision budgétaire, qui se traduisent par un véritable recul des sous-budgétisations, et l'absence de dégel de réserves de précaution. De même, le déficit, en s'établissant à 2,5 % du PIB, s'est révélé inférieur de 10 milliards d'euros à celui prévu qui était en projet de loi de finances initiale. Bien sûr, vous vous en réjouissez, monsieur le secrétaire d'État, et vous mettez en avant un progrès dans la sincérité budgétaire de l'État. Néanmoins, ce résultat est largement en trompe-l'oeil. La croissance a été de 1,7 % en 2018, en recul par rapport à l'année précédente. La consommation, principal moteur de l'activité économique, contribue moins à la croissance qu'en 2017, avec simplement 0,7 point de PIB.

Quant au déficit budgétaire, même en diminution, il est encore loin du niveau qui permettrait de stabiliser la dette, malgré une plus-value de 8,8 milliards d'euros de recettes fiscales, qui, pour l'essentiel, même si nous nous en réjouissons, ne doit rien à l'action du Gouvernement. Enfin, ce résultat est en trompe-l'oeil, car d'importantes sous-consommations de crédit en sont à l'origine. Elles concernent notamment la défense, ce qui est contraire aux engagements pris en la matière pour ce quinquennat, à la fois pour le rythme d'investissement dans nos armées et pour les modalités de financement des opérations extérieures. Elles concernent la justice, alors que ce devrait être un domaine prioritaire. Elles touchent les collectivités locales, déjà largement mises à contribution par le Gouvernement. Et ces crédits ne sont pas reportés : ils sont purement et simplement annulés Je rappellerai enfin que c'est la mission « Travail et emploi » que vous avez sacrifiée dans l'exécution budgétaire 2018, ce qui est révélateur des orientations politiques du Gouvernement. Vous avez amputé les actions dédiées à l'emploi et à la solidarité, au-delà même de ce qui était inscrit en loi de finances initiale. En 2018, vous aurez ainsi signé 90 000 contrats aidés, alors que 162 000 étaient prévus. De même que vous aurez largement sous consommé les crédits consacrés à la « garantie jeunes ». Ce sont donc bien les publics plus fragiles qui ont été sacrifiés, mais aussi les associations, les quartiers populaires, les collectivités locales, et, au total, la cohésion sociale de notre pays. La crise sociale et le mouvement des « gilets jaunes » ne trouvent pas seulement leur origine dans les mesures de votre budget initial pour 2019 ; ils découlent en premier lieu de l'exécution de votre les coups de rabot en cours d'année sont venus renforcer l'injustice de vos mesures initiales : augmentation de la contribution sociale généralisée pour les retraités, création du prélèvement forfaitaire unique, suppression de l'ISF, ces deux dernières mesures ayant coûté 3,5 milliards d'euros au budget de l'État, et ce sans toucher aux niches fiscales existantes. En guise de réforme structurelle, le budget pour 2018 et son exécution, qui a renforcé ses défauts, ont consisté à aider les grandes entreprises et les grandes fortunes- comme si elles en avaient besoin ! -et à faire porter tous les efforts par les plus fragiles, sans que le ruissellement annoncé reste autre chose qu'un mirage. Nous avons bien vu l'injustice sociale, mais nous attendons toujours l'efficacité économique et ses effets bénéfiques sur le budget de l'État.

En l'absence de modifications à l'Assemblée nationale comme au Sénat, les positions ne devraient pas varier beaucoup. Notre groupe, dans sa majorité, soutiendra de nouveau ce texte, qui est la constatation du budget exécuté l'an dernier, le premier budget à avoir été entièrement présenté, adopté et exécuté sous l'actuelle mandature. Comme en première lecture, je rappelle le constat plutôt positif : amélioration des comptes, réduction du déficit, stabilisation de l'endettement, sans toutefois recourir à une certaine « thérapie de choc », pour reprendre une expression popularisée dans les années quatre-vingt-dix, dont on aurait pu redouter les effets récessifs. Toutefois, il est peut-être trop tôt pour constater les effets de la crise des « gilets jaunes », qui se traduiront davantage lors de l'exécution du budget 2019. L'examen du projet de loi de règlement reste un moment privilégié, mais trop peu valorisé, du débat budgétaire. En effet, il permet de constater le budget exécuté l'année précédente et, ce faisant, les écarts éventuels par rapport à l'autorisation donnée en loi de finances initiale. Si les écarts d'exécution sont souvent liés aux variations non anticipées de la conjoncture- en matière de prévision économique, notre rapporteur général aime souvent à faire des comparaisons avec la météorologie -, d'autres différences sont plus révélatrices de l'engagement et du sérieux du Gouvernement. En l'occurrence, on constate effectivement le niveau plus faible des mises en réserve de crédits, ce qui traduit une meilleure anticipation des besoins de financement. De plus, l'arrêt du recours aux décrets d'avance, depuis 2017, et seulement quelques décrets d'annulation d'ampleur limitée tendent à redonner son sens et sa portée à l'autorisation parlementaire. Bien que ce ne soit pas l'objet du présent texte, on peut également saluer, dans la méthode, le retour à un véritable budget rectificatif de fin d'année, à l'image de celui qui a été présenté à l'automne dernier, et non un « second » projet de loi de finances- évolution fortement tempérée, il est vrai, par les mesures budgétaires et sociales « d'urgence », présentées en décembre.

D'autres missions connaissent également des annulations, comme la « Cohésion des territoires », principalement sur le programme « Urbanisme et amélioration de l'habitat ». Il faut remonter à 2015 pour trouver un niveau d'annulation supérieur. En crédits de paiement, les annulations sont plus limitées- moins de 1 milliard d'euros -et portent principalement sur le service de la dette, grâce en particulier à des taux d'intérêt extrêmement Toutefois, cette exécution budgétaire améliorée ne doit pas nous faire perdre de vue la situation globalement préoccupante des finances publiques. Si le taux d'endettement par rapport au PIB se stabilise, l'encours en valeur absolue continue, lui, d'augmenter. Et ce à l'heure où nombre de nos voisins sont engagés, depuis plusieurs années déjà, dans une réduction importante et continue de leur dette publique. La France se trouve dans une situation paradoxale. Avec un fort taux de dépense publique et un endettement élevé, elle tend à être comparée à des pays aujourd'hui en réelle difficulté budgétaire, comme l'Italie ou, dans une moindre mesure, l'Espagne. Mais contrairement à ces pays, qui ont été très durement touchés par les mesures de rigueur consécutives à la crise de 2010, le Gouvernement crise de 2010, le Gouvernement est globalement parvenu à maintenir notre système de protection sociale, à l'instar des pays nordiques. En cela, les troubles qui ont débuté à la fin de l'année dernière traduisent un changement de contexte important, que le Gouvernement ne doit pas sous-estimer. Je ne m'attarderai donc pas beaucoup plus sur la discussion de ce projet de loi de règlement pour 2018. Si, comme je l'ai déjà dit en première lecture, on peut constater de nettes améliorations par rapport aux années précédentes, qui justifient donc un vote favorable d'une majorité des membres de notre

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat a rejeté la loi de finances initiale pour 2018 ; le Sénat rejette aujourd'hui la loi de règlement. On peut considérer que c'est logique et respectable. Le groupe Union Centriste a choisi une autre logique : celle de la main tendue et des encouragements. Talleyrand disait : « Lorsque je me regarde, je me désole ; lorsque je me compare, je me console. » En réalité, pour les comptes publics, les comptes de l'État, c'est une double désolation. En considérant la situation financière de la France, on se désole forcément. sommes incapables de profiter des bonnes périodes, comme l'année 2018, pour essayer d'assainir nos finances publiques. Ce doit être une maladie française Le déficit augmente de 12 % en 2018 et la dette continue de progresser à plus de 2 300 milliards d'euros. Pour la rembourser, il faudrait multiplier nos impôts par sept, y compris la TVA- cela veut dire qu'il faudrait doubler le prix de tous les produits. Aucun ménage, aucune entreprise, ne pourrait supporter une telle situation. Si nous nous comparons, on se désole encore plus. Eh oui ! Le déficit baisse partout, sauf à Chypre, en Roumanie et en France.

nous voulons vous encourager, bien qu'en matière de dépenses publiques l'on observe davantage d'intentions que d'actions ... Le Premier ministre disait récemment que, pour réduire la dépense publique, toute initiative était forcément impopulaire, mais indispensable. Nous sommes d'accord,

En 2018 comme en 2017, la situation de nos finances publiques, à défaut de s'être franchement améliorée, s'est enfin stabilisée ; et, au vu de la pente sur laquelle notre pays était engagé depuis plusieurs décennies, il s'agit d'ores et déjà d'une bonne nouvelle. La crédibilité de la puissance publique envers nos concitoyens et de la France envers ses partenaires européens s'est probablement un peu renforcée : il faut le reconnaître.

Notre position sur ce projet de loi en particulier et sur la politique budgétaire en général n'a pas changé : même si nous pouvons mieux faire, sachons constater avec lucidité les progrès accomplis ces dernières années.

Nous rejoignons également la commission pour lancer une alerte à l'intention du Gouvernement, notamment pour ce qui concerne le budget de l'État. En effet, les efforts consentis sur ce périmètre sont largement insuffisants, car les baisses opérées sur les prélèvements obligatoires n'ont pas été suivies de baisses équivalentes des dépenses publiques. En conséquence, les bons résultats de 2018 tiennent plus à une conjoncture favorable qu'à l'effort structurel de réduction du déficit. C'est d'ailleurs ce que bon nombre de sénateurs reprochent au Gouvernement : ne pas profiter des temps cléments pour opérer les ajustements nécessaires. Mais il faut reconnaître qu'en France la conjoncture intérieure est souvent moins favorable, beaucoup moins favorable même, que la conjoncture extérieure : ceci explique probablement cela.

Nous le savons très bien, les fins de quinquennat ne sont jamais propices aux grandes réformes et aux économies d'envergure. Les taux d'intérêt exceptionnellement bas auxquels on prête encore à notre pays

Je rappelle que, si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble du projet de loi, dans la mesure où tous les articles qui le composent auraient été supprimés. Or, en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit sur l'ensemble du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018. En conséquence, l'article 8 va être mis aux voix par scrutin public.

Le scrutin est ouvert.

neuf articles du projet de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, le projet de loi n'est pas adopté.